et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, modifié par lettre rectificative, d'orientation des mobilités

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, ce texte présente des aspects positifs, mais également certains aspects très négatifs.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues, un Français sur quatre a déjà été contraint de refuser un emploi ou une formation en raison d'un manque de solutions de mobilité. La mobilité se trouve à la croisée de nombreuses thématiques et problématiques, qui en font un sujet si primordial : perspectives d'emploi, innovations numériques, protection de l'environnement ou encore respect des données. ans après la dernière grande loi d'organisation des transports, il était temps de revenir sur les transformations majeures affectant ce secteur et de se tourner vers les formidables opportunités qu'elles nous offrent. Une autre donnée illustre bien les enjeux sous-jacents à cette réflexion : près de quatre Français sur dix estiment n'avoir aucune alternative à la voiture. Le premier des défis est le manque de solutions de mobilité, le manque de solutions de mobilité, aujourd'hui vécu comme une source d'inégalités et d'injustices entre les citoyens comme de fractures entre les territoires. Cela donne le sentiment d'une assignation à résidence à une population sans autre réponse que la dépendance à la voiture individuelle. Le groupe Union Centriste partage pleinement les objectifs de ce projet de loi. Trente-six ans plus tard, il fallait de nouveau penser un système de mobilité qui ne soit plus un frein à l'autonomie des personnes, à la cohésion des territoires, au développement économique et au retour à l'emploi. Le groupe Union Centriste se réjouit que ce projet de loi ait d'abord été examiné en première lecture, ici, au Sénat, car les politiques de la mobilité reflètent les diversités, les spécificités ainsi que les très nombreuses opportunités de nos territoires, que nous défendons chaque jour dans cette institution.

Je le disais, le désenclavement des territoires passe par une refonte de notre système de mobilités. Si le projet de loi qui nous était présenté traduisait une approche classique par mode de transport, le Sénat a su défendre une approche multimodale Désormais, l'ensemble des territoires disposent d'une autorité organisatrice de la mobilité, contre 20 % d'entre eux auparavant. C'est assurément par une prise en compte accrue de la ruralité ainsi que des réalités territoriales que le texte s'enrichit. Désormais, l'application du mécanisme de péréquation verticale en cas de faible rendement du versement mobilité se fera par la prise en compte de la densité de la population. L'intégration de l'objectif de désenclavement à l'horizon 2025 se double de mesures concrètes visant à définir des solutions alternatives à la voiture,, par exemple, l'ouverture du transport scolaire en milieu rural l'ouverture du transport scolaire en milieu rural à des personnes âgées isolées ou fragiles, grâce à notre collègue Michèle Vullien, ou encore la possibilité de décaler les horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires pour optimiser ce transport. La deuxième priorité est en réalité une urgence : la transition énergétique. Le secteur des transports représentait 33 % de la consommation d'énergie finale en France en 2015. Il était également le principal émetteur de CO2, avec 39 % des émissions totales de gaz à effet de serre. du projet de loi, le Gouvernement semblait pourtant accepter que le transport fasse partie des secteurs qui rencontrent le plus de difficultés à atteindre les objectifs pour la croissance verte. Pour y remédier, nous saluons l'ajout aux objectifs de la programmation des infrastructures de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique ainsi que l'inscription de la diminution des émissions de gaz à effet de serre parmi les objectifs de la programmation des investissements dans les transports. Le soutien à la filière hydrogène, la possibilité donnée aux collectivités d'augmenter la taxe de séjour qui s'applique aux navires de croisière les plus polluants, ou encore la faculté accordée aux communes de créer des voies et des stationnements réservés à certains véhicules en fonction de leurs émissions de polluants sont autant de mesures pragmatiques et conformes aux ambitions de la France en matière de transition énergétique. Troisième priorité, enfin, et surtout, nous jugeons impérieux de disposer de garanties en termes de financement.

la TICPE, votée en 2014, la commission rétablit la cohérence et l'ambition de base en fléchant les recettes supplémentaires au financement des infrastructures routières et non à celui du budget de l'État. Madame la ministre, au-delà de ces trois principales priorités, nous regrettons que, par manque de pédagogie, certaines ambitions de l'avant-projet de loi, qui allaient pourtant dans le bon sens, n'aient pas été discutées au Sénat, notamment l'expérimentation de micropéages urbains. Cette mesure illustrait pourtant le passage d'une logique coercitive à une logique incitative en termes de mobilités, se traduisant par le recours aux expérimentations de nouvelles mobilités. De telles expérimentations bénéficieraient d'ailleurs pleinement d'une prise de décision décentralisée. À ce titre, nous sommes prêts à défendre un droit à la différenciation que notre pays et nos territoires attendent pour répondre aux besoins d'innovation et faire l'expérience de réformes grandeur nature. Ce n'était certes pas l'objet de ce texte, mais, alors qu'est examiné en ce moment même le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, cette question apparaît, pour le groupe comme son corollaire, qui permettrait un nouvel approfondissement de la décentralisation. Très bien ! Madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est désormais présenté est amélioré, intégrant les enjeux relatifs à la ruralité,

J'en veux pour preuve que, en donnant compétence aux présidents de département et aux préfets pour déterminer la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, nous sortons par le haut

Madame la ministre, le groupe Union Centriste votera ce projet de loi en première lecture, mais, avec le président Maurey, il tient à vous rappeler que nous attendons de votre part des précisions et des clarifications en ce qui concerne son financement. La parole est à M. Jérôme

un texte attendu par les Français et par les collectivités, tant, depuis trop longtemps, certains de nos territoires vivent mal leur isolement. La politique de la mobilité est une condition de la liberté et de l'égalité. La mobilité, c'est l'échange, qui doit être durable, effectif, et concerner tous les citoyens ; c'est également un vecteur de lien social. Nous espérons donc vivement que les dispositions de ce projet de loi permettront de donner un nouveau souffle aux transports en France, que l'on appelle aujourd'hui

nous devrons travailler. L'inscription dans le texte de l'affectation d'une fraction de la TICPE à l'Afitf permet ainsi de sécuriser les ressources de cette agence si essentielle.

ou de la nouvelle contrainte. Ne montrons pas du doigt tel ou tel secteur. L'État a besoin d'argent, les collectivités aussi. Nos territoires peuvent faire plus et ils le font déjà ; ils ont néanmoins besoin de moyens et de flexibilité. Nous nous réjouissons ainsi que la gouvernance de la mobilité ait gagné en flexibilité, en permettant une certaine adaptabilité de la compétence mobilité. Paris n'est pas la Corrèze, la baie de Somme n'est pas la région lyonnaise, une solution unique de mobilité pour l'ensemble de la France ne fonctionnera pas. Nous avons eu le souci de rendre certaines dispositions du texte plus pragmatiques et de faire davantage pour la transition écologique. Nous espérons que nos ajouts visant à promouvoir l'usage des mobilités propres et actives permettront une décarbonation des transports. La possibilité de cumuler le « forfait mobilités durables » et le remboursement d'une partie de l'abonnement de transports collectifs ne peuvent qu'encourager les salariés à recourir à des moyens de transport propres. Couvrant le vélo, le covoiturage et les véhicules électriques, ce forfait participera nécessairement à la réduction de la pollution. Nous ne pouvons cependant que regretter le fait que sa prise en charge par l'employeur n'ait pas été rendue obligatoire, comme c'est déjà le cas pour l'abonnement de transports collectifs du salarié. salarié. Nous craignons que cette prise en charge facultative ne soit appliquée que de manière réduite. La lutte contre le dérèglement climatique doit être notre priorité. Nous nous félicitons ainsi des avancées introduites en faveur du vélo

Tout au long de son examen, nous avons pu constater à quel point le texte faisait confiance aux territoires en procédant à une plus large décentralisation. C'est une bonne chose. Il fallait aussi permettre aux collectivités de réguler les moyens de transport au sein de leur bassin. effet à l'échelle locale que l'on peut le mieux apprécier les dangers de certains itinéraires et que l'on est le plus à même de poser des limites intelligentes aux nouvelles mobilités. Nous pensons que les collectivités sont les plus aptes à apporter une réponse efficace, durable et adaptée aux défis qu'elles rencontrent en matière de mobilité. À cet égard, nous nous réjouissons que le Gouvernement ait introduit la faculté, pour les régions qui le souhaitent, de se saisir de la gestion des lignes ferroviaires de dessertes fines, les fameuses petites lignes. Je pense en particulier

le texte comporte, à notre sens, de nombreuses dispositions prometteuses, pour plus de flexibilité, plus d'efficacité et plus d'écologie. Pour cet ensemble de raisons, le groupe Les Indépendants le votera. Des moyens de transport toujours plus durables, des solutions conçues au plus près des territoires et davantage de confiance aux collectivités et en nos concitoyens : voilà, mes chers collègues, ce en quoi nous croyons ! La parole

au risque de manquer d'audace, mon explication de vote aura pour objet principal de rendre compte de la position du groupe Les Républicains sur ce projet de loi d'orientation des mobilités. Pour ce faire, et là encore je vais conserver un style académique, je vais commencer par féliciter notre rapporteur, Didier Mandelli. Je profite

Je n'oublie pas non plus Françoise Gatel, rapporteur pour avis de la commission des lois, et les nombreuses améliorations dont elle et sa commission sont à l'origine en matière de gouvernance de la mobilité. Je salue enfin Benoît Huré et ses pertinentes observations sur la transposition du droit européen par ce projet de loi d'orientation des mobilités. En ce qui concerne le contenu de ce texte, les louanges adressées à notre rapporteur ne sont pas un exercice imposé.

-, qui offre, avec la programmation des investissements dans les transports, une opportunité sans précédent, pour beaucoup d'entre nous, de graver dans le marbre un projet d'infrastructure que notre terre d'élection nous réclame depuis parfois des décennies

le risque était de faire de ce projet de loi un cahier de doléances législatif avec 348 remontrances adressées au Gouvernement. Cela n'a pas été le cas. Si nos collègues de l'Ardèche ont bénéficié d'un traitement de faveur, c'est en raison de la situation unique de leur département : pas de desserte ferroviaire ou autoroutière, pas plus de route nationale non concédée à 2x2 voies ; il s'agit d'une exception en France métropolitaine. autre entorse au principe selon lequel nous ne pouvions pas nommer chacune des infrastructures indispensables au développement de nos territoires : la liaison Lyon-Turin. amendement, notre collègue Michel Savin a rappelé que la France doit honorer les accords et les traités internationaux qu'elle a signés : la convention alpine de 1991 et les traités franco-italiens de 2001, de 2012 et de 2015. La réponse du rapporteur aux nombreuses sollicitations visant à inscrire tel ou tel projet ne pouvait pas être plus équilibrée. Elle comporte deux volets : affectation intégrale de la hausse de TICPE prévue par la loi de finances pour 2015 au financement des infrastructures de transport ; consécration des projets inscrits au scénario 2 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Avant de parler des compétences, je souhaite rappeler l'engagement que vous avez pris, madame la ministre, lors de la discussion générale. Je vous cite : « pas de prise de compétence sans ressources adaptées ». justement, la faiblesse originelle d'un texte qui ambitionne de lutter contre les zones blanches de la mobilité en permettant la mise en place d'autorités organisatrices de la mobilité sur l'ensemble du territoire. Le projet est intéressant, l'intention est plus que louable,

un amendement du rapporteur, vivement souhaité par les élus locaux, doit permettre que celui-ci se fasse jusqu'au 1 juillet 2021 et non plus au 1 janvier de

! Sur les nouvelles mobilités, le Sénat a eu raison de ne pas conserver, à l'issue des travaux en séance publique, la charte facultative pour les plateformes de mise en relation. Une telle mesure n'aurait pas été conforme à ses standards en matière de qualité de la loi loi ; de plus, quel aurait été l'impact de cet OVNI législatif sur une jurisprudence en pleine effervescence ? Le Sénat ne pouvait pas cautionner ce dispositif.

suite d'une intervention de notre collègue Jean-Pierre Vial, vous nous avez assuré de l'engagement de la France à se joindre à la demande de l'Italie pour solliciter le financement à hauteur de 50 % de la part de l'Union européenne.

La parole est à M. Frédéric Marchand, pour le groupe La République En Marche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues : « Un homme est fait pour être mobile. Tout le malheur vient de l'immobilité. On use les choses en étant immobile.

Nos échanges, toujours courtois et constructifs, ont permis à ce texte, dont nous savons toutes et tous qu'il est essentiel pour notre avenir collectif, d'être sensiblement amendé et abondé.

de loi d'orientation des mobilités, que le groupe La République En Marche votera, est le résultat d'un travail collectif mené depuis maintenant plusieurs mois. Il s'agit d'abord du vôtre, madame la ministre, après des Assises de la mobilité qui ont été une vraie réussite et demeurent l'exemple d'une démarche participative achevée.

le travail de notre rapporteur, Didier Mandelli, qui a souhaité associer tous les sénateurs de notre commission ... Très bien ! ... aux nombreuses auditions organisées, permettant à celles et ceux qui le souhaitaient de s'emparer de ce formidable sujet des mobilités.

le travail de celles et ceux qui se sont succédé à la présidence de nos débats, et qui ont permis à ceux-ci de se tenir dans des conditions optimales. Oui, mes chers collègues, le Sénat a une fois de plus fait oeuvre utile s'agissant de l'épineuse question des mobilités. Il y a eu la réforme ferroviaire, il y aura désormais la loi d'orientation des mobilités : ces deux textes sont des réponses fortes à celles et ceux qui manifesteraient encore un certain scepticisme à l'égard de notre assemblée. Le Sénat fait belle oeuvre utile quand il s'empare de sujets et de textes sur le fond, et qu'il travaille sans relâche à les améliorer dans le souci de l'intérêt collectif, celui des territoires et, aussi et surtout, celui de nos concitoyens. C'est chose faite avec ce texte. Nous pouvons affirmer, sans forfanterie aucune, que la copie que nous livrons à nos collègues de l'Assemblée nationale est riche en sujets de discussion. Elle doit permettre de poursuivre la dynamique enclenchée, sans faire d'impasse sur quelque sujet que ce soit et en abordant les mobilités du quotidien sous tous les angles. Nos collègues de l'Assemblée nationale, que je salue ici, en particulier le député Jean-Marc Zulesi qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, vont pouvoir s'appuyer sur un texte ayant aujourd'hui les faveurs de nombre d'acteurs des mobilités qui ont suivi nos débats avec la plus grande attention. En effet,

de la problématique des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, des dispositions relatives à nos territoires ultramarins, de l'ouverture des données, des mobilités partagées, du développement du réseau des recharges électriques ou de la création du « forfait mobilités durables » ; et de bien d'autres sujets encore Comme toujours en pareil cas, nous pouvons nourrir des regrets de ne pas avoir été suivis par notre assemblée sur plusieurs points. C'est le cas pour le, sujet sur lequel j'ai la conviction que notre assemblée a privilégié l'émotion- légitime -d'une situation actuelle, qui n'est sans doute pas des plus satisfaisantes, au au détriment de la nécessaire concertation avec des acteurs- nous l'avons vu au fil des concertations -qui souhaitent, dans le cadre d'une régulation inéluctable du secteur, s'impliquer dans les nouvelles mobilités au service des collectivités. Je regrette aussi la frilosité de notre assemblée, qui n'a pas souhaité graver dans le marbre le respect des objectifs fixés par le plan Climat, comme la fin de la vente des véhicules essence et diesel à l'horizon 2040, la neutralité carbone du transport fluvial à l'horizon 2050, ou bien encore la réduction de 50 % des émissions de CO2 dans le transport aérien à l'horizon 2050. Je regrette que notre assemblée n'ait pas été au rendez-vous sur un sujet qui va bien au-delà des préoccupations de la jeunesse et sur lequel nous avons une impérieuse obligation d'agir et de prendre nos responsabilités, loin de toute considération partisane. Je suis persuadé que l'Assemblée nationale ne fera pas montre de la même frilosité et que cette mesure sera réintroduite. Nous avons aussi de réels motifs de satisfaction : des mesures fortes ont ainsi été prises après l'adoption d'amendements soutenus sur toutes les travées. Je me félicite de ce que la notion de mobilité inclusive se soit substituée à celle de mobilité solidaire car, ne nous y trompons pas, la question de l'inclusion des exclus dans la mobilité est une question primordiale.

Notre assemblée s'est pleinement saisie du sujet pour favoriser la pratique du vélo du quotidien, qu'il s'agisse du stationnement, de l'emport dans les trains, de l'apprentissage du vélo chez les plus jeunes, du schéma national des véloroutes ou de l'obligation de réaliser des itinéraires cyclables. Ce sont là autant de sujets sur lesquels le Sénat a fait preuve d'audace. Il ne reste plus qu'à espérer, monsieur le président, que notre assemblée se dote sous peu d'une flotte de vélos à assistance électrique pour les sénateurs et les collaborateurs : la vélo-compatibilité du Sénat sera ainsi louée partout dans l'Hexagone

Cette boîte à outils ne sera efficace qu'à la condition, ensuite, de promouvoir les expérimentations avant toute modélisation : nous avons là aussi entendu votre volonté

Le Sénat a montré la voie avec un texte qui n'a d'autre ambition que de répondre à cette préoccupation partagée par tous les élus de notre territoire, lesquels savent que tout commence par les mobilités : l'accès à l'emploi, l'éducation, la santé et la culture. Tout est enjeu de mobilité et, en votant pour ce texte, nous montrons que nous sommes à la hauteur de cet enjeu ! La parole

Conseil d'État. Nous avons d'ailleurs déposé une motion de procédure pour exprimer notre désaccord sur ces méthodes. Nous réitérons notre propos. Le Gouvernement aurait dû attendre la fin du grand débat pour tenir compte des revendications. Pour l'instant, ce qui prédomine, c'est l'inertie. Le projet de loi n'apporte aucune réponse aux enjeux soulevés, ceux de l'égal accès au service public, de la justice fiscale, du coût du transport et de la possibilité d'une transition écologique qui ne rime pas avec déclassement social pour les plus fragiles. Il ne répond pas non plus à l'enjeu défini, entre autres, par les « gilets jaunes » d'une maîtrise publique des infrastructures. Le texte ne ni de recettes nouvelles pour développer l'offre de transports collectifs. Le est maintenu sur les conditions mêmes de l'exécution du service public et de ses financements, puisque l'Afitf reste dans l'impasse, et ce malgré nos multiples propositions, comme le retour de l'écotaxe ou la modernisation du versement transport, qui n'ont trouvé aucun soutien sur ces travées. Notons tout de même la volonté du rapporteur de sanctuariser les recettes de l'Afitf grâce au fléchage d'une partie de la hausse de la TICPE. Cette fiscalité écologique, qui rapporte plus de 30 milliards pourrait cependant être davantage affectée au financement des transports, de sorte que la fiscalité écologique ne soit pas un simple alibi permettant d'alourdir les impôts de nos concitoyens. Nous ne pouvons nier certaines avancées.

va au bout de sa logique, ce projet de loi s'inscrit dans un contexte qui contredit ses objectifs. Madame la ministre, quand nous vous entendons dire que vous ne partagez pas l'idée selon laquelle le transport régulier est nécessaire sur l'ensemble du territoire, nous ne pouvons qu'être en profond désaccord avec votre vision du système de transport. Nous considérons justement que le droit au transport, qui sous-tend l'idée d'un transport public et de masse, l'idée d'un maillage du territoire en réseau, reste à développer et à conquérir pour tous. Nous considérons également qu'il convient de conserver des agents publics pour l'exécution de ces tâches si essentielles et si particulières. Pour le dire comme nous le pensons, le covoiturage, la trottinette et le vélo, qui restent des modes de transport individuels, ne font pas la maille face à l'immense enjeu des mobilités dans le cadre de flux toujours plus importants. Comprenons-nous bien, ils ont toute leur pertinence, mais dans le cadre d'une stricte complémentarité avec des modes plus structurants, notamment l'offre ferroviaire.

l'ouverture des gares par les facteurs confirme le recul du service public, tout comme la fermeture des lignes capillaires et des gares annoncée par les médias, ... Elle a raison ! ... qui conduit à la rétraction du réseau et de l'offre, comme nous l'avions prédit. La SNCF prospecte La SNCF prospecte déjà en Espagne, et les potentiels nouveaux entrants sont approchés par SNCF Réseau. Avec ce projet de loi, vous organisez le même dessein pour les transports urbains. quel est l'intérêt de la concurrence du « tous contre tous », qui permet même à la RATP de concurrencer la SNCF, et inversement, dans une logique fratricide ? d'un gâchis de temps et d'argent, alors qu'il est nécessaire de répondre à un besoin d'intérêt public. Nous considérons que la cohérence de l'offre, les logiques d'intermodalité, comme les économies d'échelle imposent de réfléchir en termes d'opérateur intégré et même- osons les mots ! -de monopole public. Au moment où les élections européennes se profilent, nous estimons qu'il faut mettre fin à ce dogme de la libéralisation à tout crin, que tous les acteurs et tous les usagers dénoncent dès lors qu'elle est mise en oeuvre. Nos gouvernements devraient non pas se comporter en petit commis de la Commission européenne, mais faire en sorte de bien réfléchir en fonction de l'intérêt de nos concitoyens. Nous pensons qu'il existe une autre voie à celle du démantèlement et de la privatisation rampante de la RATP, une autre voie que la libéralisation des transports urbains des transports urbains et de la mise en concurrence des salariés. Votre sac à dos social est un parachute percé, celui du recul des droits et des garanties pour les agents du service public La concurrence ne remplit finalement qu'une fonction, celle d'apporter une source nouvelle de profit aux acteurs privés en mal de dividendes. C'est un modèle fou qui déstructure tout ce qui fait le bien commun et qui, de ce fait, attaque les fondements de notre République. Quand nos concitoyens ne partageront plus les mêmes droits, droits, le pacte républicain sera rompu. C'est ce que vous promettez avec cette loi et vos solutions en termes de mobilités : des services publics à géométrie variable, en fonction du lieu de résidence et de la capacité contributrice de l'usager, très loin des principes d'égalité, d'adaptabilité et de continuité. Pour toutes ces raisons, auxquelles j'aurais pu ajouter la provocation faite au droit de grève et notre rejet complet du Charles-de-Gaulle Express, nous voterons contre ce projet de loi qui ne répond pas aux enjeux de mobilité, de transport et de transition énergétique. Ce texte fait fait de la route l'unique matrice de la mobilité, oubliant les enjeux liés au fret ferroviaire, « ubérisant » les acteurs et organisant le démantèlement des opérateurs et des services publics ! La parole est La parole est à M. Michel Dagbert, pour le groupe socialiste et républicain.

chers collègues, à la suite du discours prononcé par le Président de la République à Rennes en juillet 2017, nous pouvions comprendre la pause demandée en matière de grands chantiers d'infrastructures. Les gouvernements successifs avaient honoré les engagements pris au fil du temps et des majorités à l'égard des métropoles, afin de réaliser la France de la grande vitesse. Il ne faut pas le regretter, car, outre le temps gagné sur ces dessertes, c'est aussi pour la France la possibilité d'exporter un savoir-faire reconnu. Il n'en demeure pas moins que, durant la même période, c'est l'ensemble du réseau qui a pâti d'un sous-investissement. S'agissant de la route, la crise de 2008 a eu un fort impact sur l'allocation des budgets aux collectivités, conduisant à une réduction sensible de leur investissement dans le domaine l'ambition que vous portez a eu du mal à émerger au travers de ce projet de loi d'orientation des mobilités. Nous pensions sincèrement que ce texte serait une grande loi-cadre prenant en compte toutes les mobilités sans exception

De plus, votre volontarisme a été mis à l'épreuve des arbitrages de Bercy et de Matignon. Le texte présente quelques lacunes et ne nous semble pas totalement satisfaisant, notamment en ce qui concerne la question prégnante des financements. Nous regrettons à cet égard que notre proposition d'un grand emprunt n'ait pas été acceptée. Pour l'heure, il est en effet fondamental d'investir, non seulement pour entretenir et renouveler nos infrastructures, mais aussi pour accélérer la réalisation d'un bon nombre d'entre elles dans les territoires. ailleurs, la question de la contribution financière des poids lourds, notamment des poids lourds étrangers qui empruntent nos axes routiers, aurait mérité d'être traitée dans ce texte. ce texte. Notre groupe avait proposé d'instaurer une redevance kilométrique, afin de les mettre à contribution. Espérons que l'Eurovignette ne tardera pas à être mise en place. Nous nous inquiétons également des conséquences de l'ouverture à la concurrence de la RATP pour les salariés qui doivent bénéficier, selon l'expression consacrée, d'un « sac à dos social ». Encore faut-il en vérifier le contenu ! Nous y serons attentifs.

Au-delà de ces points, c'est avec une certaine gourmandise que le Sénat s'est attelé à la tâche, notamment sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont je veux saluer le président, ainsi que le rapporteur, notre collègue Didier

tous légitimes, pour défendre, ici, un tronçon d'autoroutes, là, une voie de chemin de fer, ailleurs, la modernisation d'une écluse. Pour autant, le travail de nos collègues a permis un certain nombre d'avancées, sur lesquelles je veux rapidement revenir. Ainsi, le Conseil d'orientation des infrastructures est pérennisé. La La proposition émise par notre groupe en commission concernant le transfert de la gestion de certaines lignes ferroviaires nationales aux régions a également été intégrée au texte. La sanctuarisation des ressources de l'Afitf avec l'affectation de l'intégralité du produit de la hausse de la TICPE est aussi à saluer.

Il est agréable de noter la prise en compte des spécificités et des enjeux portés par nos collègues ultramarins sur les problématiques maritimes et de continuité territoriale. Nous nous réjouissons également de la consécration comme une priorité de la nécessité de développer le transport fluvial et de mener une politique volontariste en la matière, l'inscription du canal Seine-Nord Europe dans la loi ne lève pas les incertitudes liées à son financement. Nous avons accueilli avec satisfaction les propos du Président de la République devant les élus des Hauts-de-France vendredi dernier.

ce texte a pu susciter une certaine forme de déception chez ceux qui attendaient une véritable révolution dans le domaine. Néanmoins, force est de constater que nous sommes nombreux à saluer les avancées de ce texte, en particulier son orientation stratégique qui permet de mettre enfin l'accent sur les mobilités du quotidien, grâce notamment au rôle renforcé des collectivités locales. Nous sommes aussi nombreux à saluer l'esprit d'ouverture du Gouvernement, ainsi que la prise en compte des attentes des différents groupes par le rapporteur. À la lecture du projet de loi, un double enjeu apparaît très clairement : celui de désenclaver le territoire, tout en luttant contre la pollution liée aux transports ; ces deux objectifs ne sont pas contradictoires si l'on sait s'en donner les moyens. Je ne peux pas entamer mon intervention sans évoquer la forte hausse du nombre des morts sur les routes depuis le début de l'année. Cette augmentation particulièrement inquiétante nous rappelle que toute politique de prévention doit s'accompagner d'une politique de répression efficace. La dégradation des radars automatiques au cours des derniers mois a entraîné une baisse de la vigilance, qui doit inciter les pouvoirs publics à agir rapidement. Début mars, 75 % des radars étaient encore endommagés

Depuis la présentation de ce projet de loi, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l'instabilité du financement de l'Afitf, en raison notamment de l'instabilité du produit des amendes-radars. Il manque des centaines de millions d'euros à l'Agence pour qu'elle puisse mener à bien ses projets et concrétiser l'ambitieux plan d'investissement de l'État en la matière. Certes, un cap clair un cap clair et innovant est fixé, mais comment s'en réjouir tant que l'on ignore comment il sera financé ? C'est pourquoi, considérant qu'il fallait être à la hauteur des enjeux, les sénateurs ont fait le choix d'inscrire dans la loi des ressources pérennes et sanctuarisées pour l'Afitf. Nous espérons que cette position sera partagée par nos collègues de l'Assemblée nationale. Nous attendons aussi beaucoup du Gouvernement, qui nous promet des solutions issues du grand débat dans le prochain projet de loi de finances.

Madame la ministre, vous avez porté l'ambition de couvrir 100 % du territoire en autorités organisatrices de la mobilité, en affirmant qu'il n'y aurait pas de transfert de compétences sans ressources adaptées. Vous renvoyez sur ce point à la prochaine grande réforme de la fiscalité locale.

une fracture qui divise la France des métropoles et la France des territoires, délaissée, abandonnée, menacée par des décennies de sous-investissement. Une politique centrée autour des bassins de mobilité et des élus locaux permettra certainement de pallier certaines défaillances actuelles. La décentralisation renforcée, que nous appelons tous de nos voeux, prend forme peu à peu. Elle nécessite néanmoins, comme l'a très justement rappelé notre collègue Ronan Dantec, une forte péréquation et une solidarité nationale assumée. Hors des grandes agglomérations, la voiture demeure indispensable. À l'échelle du pays, la voiture reste même le mode de déplacement domicile-travail de plus de 70 % des actifs.

de renforcer le maillage territorial des lignes ferroviaires, qui apparaît comme une étape indispensable à l'émergence d'une mobilité du quotidien moins dépendante de la voiture. Ces petites lignes qui structurent l'espace doivent absolument être préservées et seront, j'en suis sûr, l'un des maillons essentiels de la mobilité de demain. Nous saluons à ce titre l'adoption d'un amendement, soutenu notamment par notre groupe, qui permet la gestion de certaines lignes par les régions qui en feraient la demande. Je me réjouis aussi de l'adoption d'un amendement permettant d'inscrire une possibilité de concomitance des travaux de modernisation et de régénération sur les lignes d'équilibre du territoire, trop longtemps délaissées et pour lesquelles le temps de parcours s'est beaucoup allongé en trente ans, mais qui restent tout aussi primordiales pour la mobilité et le désenclavement. Nous aurions toutefois souhaité voir émerger des engagements plus fermes en ce qui concerne la vente des véhicules thermiques neufs. Près de 94 % des voitures présentes sur le territoire fonctionnent encore avec un moteur thermique. La marge de progression est immense : elle doit inciter l'État et les parlementaires à s'engager de manière plus énergique. Si nous voulons la fin des véhicules thermiques en 2040 et la neutralité carbone en 2050, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Malgré une délivrance soumise au bon vouloir de l'employeur, le « forfait mobilités durables » donne un premier signal positif aux usagers en les incitant financièrement à opter pour des modes de transport moins polluants.

le rehaussement de la part minimale de véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules d'entreprise, ainsi que des mesures visant à réduire la pollution des navires. Sur proposition du RDSE, le Sénat a également souhaité étendre à tous les territoires la possibilité de créer des zones à faibles émissions. Pour des raisons prioritaires de santé publique, il était important de supprimer le seuil initial de 100 000 habitants. Puisqu'il est question de santé publique, j'aimerais achever mon propos en saluant les mesures importantes qui ont été prises en faveur du vélo, même si ce mode de déplacement ne peut pas être utilisé partout avec la même facilité. Associées au grand plan mis en place par le Gouvernement, elles permettront de renforcer la place de ce mode de transport vertueux, à la fois pour l'environnement et pour la santé. Vous l'aurez compris, le groupe du RDSE salue les avancées portées par ce projet de loi, notamment les 23 amendements qu'il a fait adopter et qui reprennent pour partie des mesures contenues dans la proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires. Nous voterons donc à la quasi-unanimité en faveur de ce texte, largement enrichi par le Sénat. Mes chers aura lieu en salle des conférences. Je remercie nos collègues Yves Daudigny, Guy-Dominique Kennel et Patricia Schillinger, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Je rappelle qu'une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais saluer l'adoption, par une très large majorité, du projet de loi d'orientation des mobilités et vous redire ma conviction que ce texte est essentiel pour répondre aux fractures territoriales et sociales, qui minent notre pays, et aux difficultés exprimées par nombre de nos concitoyens, notamment dans le cadre du grand débat. Ce projet de loi apportera des réponses concrètes aux besoins actuels et à venir en matière de mobilité du quotidien. La rédaction issue de vos travaux en première lecture respecte les grands équilibres que j'ai défendus. Je ne peux que m'en réjouir. Je me félicite notamment du consensus existant sur l'un des principes structurants du texte, à savoir la couverture complète du territoire par des autorités organisatrices chargées de la mobilité. Cette mesure peut paraître technique, mais c'est grâce à elle que plus aucun Français ne sera laissé demain sans solution. Je note également l'intérêt fort du Sénat pour les mobilités actives, en particulier le vélo, et plus largement pour les enjeux de transition énergétique qui se posent pour tous les modes de transport. Enfin, concernant la programmation des infrastructures, je me réjouis que vous partagiez la priorité donnée aux transports du quotidien et je remercie le Sénat d'avoir respecté l'économie générale de cette programmation, même si- j'ai eu l'occasion de le dire -je ne souhaitais pas que ce titre soit placé en tête du texte. Un certain nombre de sujets devront être approfondis à l'Assemblée nationale, notamment la question du financement, du ou de la billettique, mais je voudrais me féliciter de nouveau de la richesse des débats qui ont eu lieu durant cet examen et, malgré quelques divergences, saluer le rôle constructif et la mobilisation de votre Haute Assemblée pour enrichir ce texte. Mes chers

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019. La parole est à Mme la secrétaire d'État, à qui je souhaite la bienvenue au Sénat.

pour porter au mieux les questions européennes dans ces heures agitées. Je suis aussi très heureuse de pouvoir vous rencontrer dans le cadre de ce nouveau format de débat, postérieur au Conseil européen. J'espère que cela permettra des échanges riches, après un Conseil européen qui a été particulièrement commenté.

Le Conseil européen a effectivement été dominé par le retrait britannique et la demande de Mme May de reporter la sortie jusqu'au 30 juin. Je ne reviens que rapidement sur le résultat, que vous connaissez. Sous l'impulsion du Président de la République, un accord a été trouvé, avec deux options pour cette extension

en l'absence de soutien de la Chambre à l'accord de retrait. Pourquoi le 12 avril ? C'est la date limite pour que Londres décide d'organiser des élections européennes afin de disposer de députés au Parlement européen, comme ceux que la France y enverra à la suite des élections du 26 mai prochain. Il se trouve que la Chambre des communes a rejeté une troisième fois, le 29 mars, l'accord de retrait. Il a manqué 58 voix à Mme May, un nombre en nette réduction, puisqu'il lui en manquait 149 le 12 mars et 230 le 16 janvier. Pour autant, nous savons, dans cette assemblée comme dans d'autres,

qu'il y a un risque à voir passer une solution à leurs yeux bien pire que l'accord de retrait, comme une union douanière permanente, laquelle n'a échoué que de 3 voix hier soir. Dans ce cas, l'accord de retrait peut finalement faire l'objet d'un vote favorable avant le sommet européen du 10 avril. Une brève extension technique supplémentaire serait alors nécessaire pour permettre la ratification. Ce scénario reste peu probable au vu des derniers mouvements à la Chambre, mais n'est pas impossible. Ce serait la meilleure solution.

Des recrutements ont été lancés, la construction des infrastructures est en voie d'achèvement et des campagnes de tests pour l'exercice des différents contrôles sont en cours. Nous sommes donc prêts s'il faut nous

Cette hypothèse devrait par ailleurs être soigneusement encadrée afin que le Royaume-Uni soit traité comme un État membre pas tout à fait comme les autres

Nous sommes donc toujours dans une période très incertaine. Il revient au Royaume-Uni de faire ses propres choix- des votes ont de nouveau lieu au Parlement demain et, aujourd'hui, se tiennent des réunions du cabinet extrêmement importantes. Il est clair que l'Union européenne doit continuer à manifester son unité et sa détermination à défendre les intérêts des Européens, notamment, comme le répète Michel Barnier, notre négociateur,

Ces discussions sur le retrait du Royaume-Uni ne doivent pas nous faire perdre de vue notre objectif central de relance du projet européen. L'ordre du jour du Conseil européen des 21 et 22 mars nous a permis, et c'est heureux, de présenter plusieurs des idées exposées par le Président de la République dans sa tribune pour une renaissance européenne pour défendre notre liberté, protéger notre continent et retrouver l'esprit de progrès.

Les chefs d'État et de gouvernement ont abordé tant l'avenir du marché intérieur que les politiques qui y sont liées, notamment l'économie numérique, la politique industrielle et, bien sûr, la recherche et l'innovation. En particulier, le Conseil européen a engagé une discussion sur la nécessité d'une véritable politique industrielle européenne. Comme nous le souhaitions, le Conseil européen a invité la Commission à présenter, dès la fin de 2019, une vision stratégique de long terme sur l'avenir de l'industrie européenne, soutenue par des mesures concrètes. Conformément aux propositions formulées par la France et l'Allemagne, cette stratégie devra en particulier soutenir les nouvelles technologies et s'assurer des financements nécessaires, notamment en ayant recours au Conseil européen de l'innovation.

La Commission doit étudier d'ici à la fin de l'année les évolutions nécessaires pour répondre aux défis des évolutions technologiques et de la concurrence mondiale. L'enjeu est de mieux défendre nos technologies, nos entreprises et nos marchés,

en particulier sur le scénario de neutralité carbone en 2050, que nous souhaitons voir adopter dans la perspective du sommet Action climat de l'ONU en septembre 2019. Comme le Président de la République l'a souligné, les conclusions du Conseil européen sur le climat sont décevantes. Alors que les

Renouer avec l'esprit de progrès qui caractérise le projet européen, c'est aussi, comme le propose le Président de la République, créer une banque européenne du climat pour mieux financer la transition énergétique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est enfin se fixer des objectifs ambitieux concernant le cadre financier pluriannuel, dont l'objectif de dépenses en faveur du climat doit être revu à la hausse par rapport à la proposition de la Commission. Troisième sujet, les conclusions du Conseil européen font également état et la nécessité de protéger l'intégrité démocratique des élections européennes et nationales dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce sont des enjeux essentiels pour notre liberté démocratique. Le Président de la République a ainsi proposé que des experts européens puissent être déployés immédiatement en cas de cyberattaques ou de campagnes de désinformation. Dans le prolongement des derniers rapports publiés par la Commission, le 20 mars, sur les progrès réalisés par les plateformes en ligne, les conclusions du Conseil européen appellent ces plateformes à renforcer leurs efforts dans la mise en oeuvre du code de bonnes pratiques contre la désinformation et à garantir des normes plus élevées de responsabilité et de transparence. Quatrième sujet, nous restons nous restons déterminés à oeuvrer pour renforcer la convergence économique et sociale au sein de l'Union, qui est au coeur du projet européen, pour nous doter de ce que le Président de la République appelle un « bouclier social ». C'est le sens de l'action que nous avons menée avec la création d'une autorité européenne du travail, ou encore de nos efforts pour lier solidarité financière et convergence sociale dans le prochain budget européen. Les chefs d'État et de gouvernement reviendront sur tous ces sujets- hormis, du Brexit -lors du sommet informel de Sibiu le 9 mai prochain, puis à l'occasion de l'adoption, en juin prochain, du programme stratégique pour la période 2019-2024, qui fixera les orientations et priorités politiques pour le prochain cycle institutionnel. Sur la méthode, nous voulons nous appuyer, pour définir les priorités de l'Union, sur les principales préoccupations et attentes des citoyens, telles qu'elles ont été exprimées, en France et au-delà, dans les consultations citoyennes sur l'Europe qui se sont tenues au second semestre de 2018, et sur une conférence sur l'Europe, qui réunira tous les acteurs nécessaires d'ici à la fin de l'année, pour définir les changements nécessaires à mettre en oeuvre. Au fond, en France, nous avons eu le grand débat national ; en Europe, les consultations citoyennes sont également là pour alimenter cette feuille de route stratégique 2019-2024, pour s'assurer que l'Europe parle bien des préoccupations concrètes des citoyens à travers l'Union. Dernier point pour conclure : le Conseil européen a échangé sur les relations avec la Chine afin de préparer le sommet Union européenne-Chine du 9 avril. La discussion La discussion a donné lieu à un constat largement partagé sur le fait que la Chine est à la fois un partenaire et un concurrent pour l'Union européenne. Il est essentiel que les Vingt-Sept restent unis et défendent leurs intérêts économiques et stratégiques face à la Chine. L'Union doit être ferme et exiger de la réciprocité, notamment dans l'accès aux marchés. Le Président de la République a résumé les discussions en estimant que, malgré certaines divergences de vue, « le temps de la naïveté de l'Union envers la Chine était révolu

La signature par le vice-Premier ministre italien et les autorités chinoises d'un accord de participation au projet des nouvelles routes de la soie souligne à quel point il est indispensable de renforcer encore davantage la coopération européenne dans ce domaine avant le sommet « 16+1 » du 12 avril en Croatie. je vous remercie de votre accueil et je me réjouis maintenant d'entendre vos commentaires et vos questions.

et de mener une action résolue pour la relance du projet européen, qui reste notre priorité absolue. En traitant de sujets aussi divers que le Brexit, la Chine ou encore la compétitivité, le dernier Conseil européen a porté, au fond, sur la capacité de l'Europe à préserver son unité et à jouer un rôle, à l'avenir, au sein du concert des grandes puissances. L'Union européenne, hélas ! se fragmente ; elle concentre une grande partie de son énergie sur la gestion du Brexit, alors que des défis immenses l'attendent si elle veut préserver son modèle économique et social, ses valeurs et sa capacité à être un acteur qui compte dans les relations internationales. les relations internationales. Le Brexit, tout d'abord. Deux ans après le début des négociations, le scénario catastrophe se poursuit, avec les trois hypothèses que vous venez d'évoquer. Pour la troisième fois consécutive, le Parlement britannique a rejeté l'accord de retrait. Nous attendons la date fatidique du 12 avril- dans dix jours -avant laquelle le Royaume-Uni doit proposer une alternative ou se résigner à un, une sortie brutale de l'Union européenne. L'Union européenne a souhaité que le Royaume-Uni reste maître de son destin, mais nous subirons tous les conséquences de ses choix. Sur la période 2016-2018, la décision du peuple britannique a déjà fait perdre, mes chers collègues, 6 milliards d'euros aux exportateurs français La dépréciation de la livre, le ralentissement de la croissance outre-Manche créent des conditions défavorables qui, malheureusement, vont perdurer. Sur le plan géostratégique, le Brexit est une aberration. C'est pourquoi nous devrons nous atteler, au cours des prochains mois, à repenser les cadres de la sécurité et de la défense européennes. La dynamique positive observée dans ce domaine depuis quelques années reste néanmoins à confirmer. Le Royaume-Uni doit pouvoir conserver le rôle essentiel qui est le sien dans l'architecture de sécurité et de défense de l'Europe. La Chine, ensuite. L'Union européenne semble prendre timidement conscience de l'ampleur des défis posés par la Chine, ce qui n'a malheureusement pas empêché l'Italie de se démarquer de ses partenaires en signant un accord bilatéral avec Pékin. L'unité dont l'Europe devrait pouvoir se prévaloir face à la Chine est mise à mal. Nous le regrettons.

alors que la France y maintient difficilement 1 400 militaires, malgré notre position historique. La Chine investit massivement dans des infrastructures civiles et militaires, en échange d'un endettement massif- et donc de dépendance -de ces pays. C'est une stratégie qu'elle démultiplie à l'envi, invoquant souvent le multilatéralisme, comme le président Xi Jinping l'a fait, ici même, au Sénat, alors qu'elle privilégie, en réalité, des relations bilatérales systématiquement déséquilibrées en sa faveur. La compétitivité économique de l'Europe, L'époque où l'Union européenne avait pour vocation principale de décloisonner le continent pour créer un grand marché est, hélas ! dépassée. L'Union européenne et les nations qui la composent doivent aujourd'hui assumer collectivement leur place de deuxième puissance économique mondiale. Il faut donc aider nos entreprises à se projeter au niveau international, et non pas les affaiblir en leur appliquant des règles obsolètes. L'émergence de grands champions européens dans les domaines technologiques d'avenir est un impératif stratégique. L'échec de la fusion d'Alstom et Siemens doit nous servir de leçon pour réformer l'Union européenne. Face aux grandes puissances économiques que sont la Chine et les États-Unis, la naïveté de l'Europe n'a que trop duré. Elle ne pourra résister et éviter le décrochage qu'en surmontant ses divisions et en regroupant ses forces. C'est dire l'importance de la tâche qui attend l'Union européenne et ses États membres, après l'élection du prochain Parlement européen. Madame la secrétaire d'État, nous le voyons bien, l'Europe est à un tournant de son histoire. Puissiez-vous parler au nom de la France pour faire prévaloir nos intérêts, mais aussi pour préserver les valeurs d'une Europe qui réponde vraiment aux aspirations de nos concitoyens ! La parole

Plusieurs sujets intéressant la commission des finances ont pu toutefois être abordés à l'occasion du Conseil européen du mois de mars. Tout d'abord, celui-ci a approuvé les recommandations du Conseil sur la politique économique de la zone euro dans le cadre du semestre européen.

Dans le cadre du semestre européen, le Gouvernement devrait nous communiquer sous quinzaine le programme de stabilité et le programme national de réformes, qui feront l'objet d'un débat en séance publique.

Ensuite, pour renouer durablement avec la croissance, le Conseil européen a insisté sur le nécessaire renforcement du marché unique, invitant la Commission européenne à présenter un plan d'action d'ici à 2020. Dans ses conclusions, le Conseil européen a lié la nécessité de supprimer les verrous du marché unique et celle d'aboutir à une fiscalité juste, appliquée au sein de l'Union européenne. Sur ce dernier point, au-delà des simples déclarations d'intention, force est de constater que la plupart des dossiers fiscaux sont bloqués au Conseil. Je pense notamment à l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés.

compris au plus haut niveau, avancent l'idée d'une TVA à taux zéro, alors que c'est strictement impossible, sauf à y revenir par la règle de l'unanimité. Certaines mesures sont carrément enterrées. Je pense notamment à la taxation des services numériques au niveau européen. S'il est donc ambitieux, l'agenda de la Commission européenne s'annonce toutefois délicat à mettre en oeuvre pour aboutir à des mesures concrètes. Par ailleurs, le Conseil européen a posé les jalons du mandat de la prochaine Commission européenne en matière de compétitivité et de politique commerciale. En effet, après l'échec de la fusion entre Siemens et Alstom, les États membres questionnent les fondements du droit européen de la concurrence au regard des ambitions industrielles de l'Union européenne. Le Conseil européen a ainsi invité la Commission à présenter des « actions concrètes » d'ici à la fin de l'année, même si les ingrédients de la concurrence européenne demeurent : concurrence loyale, mais aussi protection des consommateurs et des intérêts stratégiques de long terme de l'Union européenne. En matière de politique commerciale, le Conseil européen a proposé de relancer les discussions sur la réciprocité de l'ouverture des marchés publics. L'unité des États membres sur cette question semble toutefois mise à l'épreuve, comme le prouve l'adhésion de l'Italie au projet des « nouvelles routes de la soie » avec la Chine. Enfin, l'interminable épisode du

regret, à une sortie possible sans accord. Le Brexit conduirait à une perte pour le budget de l'Union européenne, si le Royaume-Uni ne respectait pas son engagement de s'acquitter des 50 milliards d'euros

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, m'a fait l'honneur de me confier le soin d'introduire, au nom de la commission, ce débat consécutif au Conseil européen des 21 et 22 mars dernier et de vous souhaiter, madame la secrétaire d'État, le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. À une semaine de la date annoncée du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce Conseil européen a consacré plus de temps que prévu à ce sujet majeur. Mais, c'est heureux, le Brexit n'a pas entièrement occulté les autres questions stratégiques à l'ordre du jour : l'approche européenne face à la Chine et la situation économique de l'Union. Concernant le Brexit, la demande de son report est arrivée très tard. Saisi la veille par Mme May d'une demande d'extension de l'article 50 jusqu'au 30 juin, le Conseil européen a réagi vite et bien : la solution retenue, qui concède une extension jusqu'au 22 mai en cas d'approbation de l'accord de retrait par la Chambre des communes, et seulement jusqu'au 12 avril dans le cas contraire, est dans l'intérêt de l'Union européenne. Ce séquençage protège en effet le scrutin européen, ouvert du 23 au 26 mai, des risques juridiques inhérents à sa tenue au Royaume-Uni, obligatoire tant que ce pays reste membre de l'Union. En outre, cette dernière ne prend pas la responsabilité du choix de l'issue, mais la renvoie très opportunément au Royaume-Uni : celui-ci est tenu de se positionner avant le 12 avril, car, au-delà, il ne serait plus en mesure d'organiser les élections européennes. Ce dispositif, d'inspiration française dit-on, apparaît bien conçu, même si la situation reste confuse à ce jour, avec le troisième refus de l'accord de retrait, intervenu vendredi dernier au Parlement britannique. Deuxième motif de satisfaction : le front uni que le Conseil européen a affiché face à la Chine, à l'approche du sommet Union européenne-Chine prévu dans une semaine. semblent prendre progressivement conscience de la nécessité de s'accorder sur la ligne à tenir face à la Chine, à la fois partenaire, concurrent économique et rival systémique. Le Conseil européen a notamment fait valoir la nécessité de parvenir à un accord sur l'instrument garantissant une réciprocité dans l'accès aux marchés publics : finissons-en avec la naïveté de l'Union européenne, laquelle ouvre ses marchés à des États qui verrouillent les leurs Le Président de la République a tenu à conforter l'image d'une Europe unie face à la Chine, en invitant à ses côtés le Président Juncker et la Chancelière Mme Merkel à Paris, où était reçu le Président chinois mardi dernier. Après les accrocs franco-allemands par voie de presse, cette démarche nous a paru salutaire, mais l'unité est fragile. La récente signature d'un mémorandum d'entente entre la Chine et l'Italie sur les nouvelles routes de la soie en est la preuve. La crainte exprimée par plusieurs États membres de se priver du bénéfice des investissements chinois en est une autre. Le prochain sommet en format « 16+1 », entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, risquait d'en apporter une troisième preuve il a donc été convenu de se conformer aux décisions issues du sommet Union européenne-Chine, qui se tiendra juste avant. Il y a là sans nul doute un progrès, mais la vigilance reste de mise. l'approche européenne concertée pour assurer la sécurité des réseaux 5G sera un prochain test. Dernier sujet traité par le Conseil européen : la situation économique de l'Union européenne. Le Conseil européen a conclu à la nécessité d'asseoir le rôle de l'Europe sur la scène économique mondiale par cinq leviers : l'Union économique et monétaire, le marché unique, la politique industrielle, la politique numérique et la politique commerciale. En outre, le numérique et l'intelligence artificielle sont reconnus comme des priorités. Cette approche intégrée préfigure une stratégie qui pourrait enfin transformer l'Union en puissance. C'est notre principal motif de satisfaction après ce Conseil européen, qui n'aura finalement

pour votre nomination, comme l'ont fait mes collègues. Il est difficile, cet après-midi, d'échapper au Brexit. Je me limiterai à quelques observations rapides.

et l'efficacité des mesures, d'autant qu'une frontière a, par définition, pour caractéristique d'être gérée à deux. Nous ne pourrons être prêts pour ce rendez-vous que si nos homologues britanniques le sont également. Vous savez aussi, madame la secrétaire le degré de préparation de nos entreprises reste aussi en discussion. Nombre d'entre elles ont d'ailleurs perdu légitimement- c'était une réussite de l'Union européenne -les savoir-faire liés à la gestion des frontières douanières. Deuxièmement, le modèle parlementaire britannique souffre, alors que son ancienneté et sa solidité ont fait notre admiration, ainsi que celle des pères de notre Constitution. Les commentaires sévères sur nos collègues britanniques abondent. Je ne les partage pas. D'une part, leurs difficultés montrent la force, la pertinence de ce qui a été bâti au cours des décennies par et avec l'Union européenne. D'autre part, partout en Europe, et pas simplement au Royaume-Uni, il est devenu difficile de passer des accords, de faire des concessions, de trouver des compromis. Cette idée selon laquelle le peuple souverain aurait une réponse simple à des questions complexes et que seule la déconnexion de la démocratie représentative ne lui permettrait pas de prendre les bonnes décisions est, vous le savez, ravageuse, des États-Unis à l'ensemble de l'Europe. Nos propres difficultés, mes chers collègues, à mettre fin à la crise des « gilets jaunes à mener nos arbitrages, à trouver des accords qui puissent être acceptés par toutes les parties de notre « archipel social »- si vous me permettez cette formule -démontrent qu'un modèle européen historique de prise de décision est attaqué. Exprimé autrement : les difficultés des Britanniques sont le reflet de nos propres difficultés, et réciproquement. Troisièmement, le Brexit vampirise la réflexion, l'énergie et l'action de l'Union européenne. Nous avons à préparer un nouveau mandat européen, une nouvelle Commission, nous avons relancé une dynamique européenne, une Europe de la souveraineté partagée.

d'élargir le regard et que vous ayez indiqué que le travail continuait pendant le Brexit avec l'avenir du marché unique, avec les questions d'orientation stratégique sur le climat ou les progrès dans la lutte contre la désinformation. Vous avez mis également en perspective

tel un feuilleton qui n'en finirait pas, les rebondissements se sont succédé depuis le Conseil européen des 21 et 22 mars dernier sur des sujets pourtant essentiels pour l'Union européenne. tout d'abord, et surtout : le Brexit. Les Européens n'ont pas cédé aux pressions britanniques et ont décidé de remettre la balle dans le camp de Theresa May alors qu'elle demandait un report au 30 juin.

Les parlementaires britanniques en ont, pourtant, décidé tout autrement en reprenant la main avec une série de votes indicatifs sur la forme que doit prendre le Brexit, votes qui n'ont rien donné et qui conduisent de plus en plus à ce qui ressemble à une voie sans issue, allant jusqu'à la démission désespérée de Theresa May ! Mais qui pour la remplacer ? Nous ne le savons pas. Permettez-moi de commencer à douter du comportement de ces élus qui n'agissent pas à la hauteur de leurs responsabilités, en mettant en danger leur pays, leurs concitoyens, leurs entreprises, mais aussi leurs partenaires historiques et économiques. Repousser la date du Brexit, sans véritable raison et sans explication donnée aux citoyens européens, n'enverra pas un bon signal et risque, au contraire, de renforcer les sentiments d'éloignement et d'incompréhension tant décriés par certains. À quelques semaines d'une échéance électorale primordiale pour l'Europe, cela ne peut être accepté. Les 27 États membres sont et doivent rester plus que jamais fermes et unis face à cette situation édifiante. L'Europe doit garder la main sur ce calendrier pour qu'il ne vienne pas perturber la bonne tenue de la campagne des élections européennes, mais également l'installation du futur Parlement européen, qui aura beaucoup à faire pour l'avenir de nos territoires. C'est maintenant aux dirigeants britanniques de s'expliquer devant leurs citoyens et électeurs. La décision du Conseil européen est donc une façon de mettre le Royaume-Uni devant ses responsabilités et doit, même si nous pouvons le regretter, s'appliquer le 12 avril en cas de. Deuxième point : les décisions concernant les relations de l'Union européenne avec la Chine, qu'il convient de saluer. J'avais alerté Nathalie Loiseau à ce sujet lors de notre débat préalable au Conseil européen et il semble que les États membres aient pris la mesure de l'urgence de faire front uni face à cette puissance économique mondiale. Sans céder aux sirènes du protectionnisme, le Conseil européen a décidé de multiplier les mécanismes pour répondre à la concurrence étrangère jugée déloyale. C'est un sujet stratégique fondamental pour les États membres européens, qui doivent plus que jamais parler d'une seule voix. C'est chose faite puisque le premier acte concret de cette nouvelle politique pourrait être l'adoption d'un nouvel instrument destiné à assurer la réciprocité entre l'Union européenne et la Chine dans l'attribution des marchés publics. Il s'agit là d'un enjeu considérable puisque ces derniers pèsent 2 400 milliards d'euros, soit plus de 16 % du produit Cela s'est aussi traduit, très rapidement, dans les faits, lors de la visite du Président chinois Xi Jinping la semaine dernière en France, accueilli par un front uni composé de la France, de l'Allemagne et de la Commission européenne. C'est cette politique coordonnée et unie entre les États membres qui doit prévaloir face à des intérêts politiques de court terme. L'Europe devra rester vigilante et passer les mêmes messages lors du sommet Union européenne-Chine le 9 avril prochain. Troisième point : la lutte contre la désinformation. Je note l'appel du Conseil pour renforcer les efforts coordonnés visant à s'attaquer aux aspects intérieurs et extérieurs de la désinformation et à protéger les élections européennes et nationales dans l'ensemble de l'Union européenne. Le renforcement de sa résilience face aux menaces extérieures est essentiel. Les élections européennes en seront le prochain test, et j'espère qu'il sera positif. enfin : même si beaucoup reste à faire, je salue les conclusions du Conseil visant à mettre en place une véritable politique industrielle européenne. Je serai attentive au document que présentera la Commission européenne d'ici à la fin de l'année concernant sa vision à long terme pour l'avenir industriel de l'Union européenne et les mesures concrètes assorties, destinées à la mettre en oeuvre. Des pistes pour une politique industrielle modernisée ont d'ailleurs déjà été présentées par un groupe de réflexion interne à la Commission, en misant notamment sur le soutien aux projets de technologies avancées et la protection des entreprises européennes. Il faudra s'en inspirer. Il semblerait aussi opportun de réfléchir à la pertinence d'une révision de la politique européenne de concurrence pour que des situations comme celle que nous avons connue avec Alstom et Siemens ne se reproduisent plus. Un nouvel équilibre doit être trouvé entre ouverture et protection du marché européen. Ces décisions du Conseil européen des 21 et 22 mars dernier sont donc stratégiques pour l'avenir de l'Union européenne, pour maintenir sa cohérence et pour la protéger au mieux des potentielles menaces extérieures. Gageons que les engagements pris seront suivis d'effets concrets. La parole est à M.

je me réjouis de la tenue de ce débat européen en séance publique, qui tombe à point nommé. Il nous donne l'occasion de nous exprimer non seulement sur les conclusions du dernier Conseil européen, mais aussi sur les récents rebondissements intervenus dans le « feuilleton » du Brexit. J'axerai mon propos sur trois dossiers en particulier, qui mettent à rude épreuve l'intégrité et la force du projet européen : le Brexit, bien sûr, les relations entre la Chine et l'Union européenne, ainsi que les enjeux de cybersécurité.

Cet accord est venu proroger la date de sortie effective, tout en préservant une unité infaillible entre les États membres. Il a réaffirmé notre position constante selon laquelle l'accord de retrait ordonné n'est pas renégociable.

et je ne suis pas sûr que nous arrivions au résultat final espéré. Plus marquant encore, le Parlement britannique n'est pas non plus parvenu à se mettre d'accord sur les huit options alternatives de retrait qui avaient été proposées par des parlementaires. Par la force des choses, le débat de ce jour est devenu un débat préalable au Conseil européen extraordinaire du 10 avril prochain, qui a été convoqué par le Président du Conseil européen, Donald Tusk, en vue d'anticiper la nouvelle date fatidique du 12 avril. Le scénario du pire, qui implique la concrétisation d'un, semble plus que jamais possible. Dans une communication faite le 25 mars, la Commission européenne a indiqué avoir finalisé ses préparatifs d'un Brexit sans accord. Fort heureusement, même si tout n'est pas achevé, le gouvernement français s'est aussi préparé suffisamment tôt à cette hypothèse. Une dernière ordonnance prise sur le fondement de la loi relative aux mesures de préparation au Brexit a été présentée en Conseil des ministres le 27 mars dernier. S'en est ensuivie la publication de trois décrets et d'un arrêté, qui permettent d'avancer. Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous dire si l'ensemble des mesures législatives et réglementaires ont été prises ? Comment jugez-vous désormais le niveau de préparation de nos entreprises françaises à un ? Notre pays estime que « l'idée d'une extension longue, impliquant une participation du Royaume-Uni aux élections européennes, ne pourra être examinée que si le plan alternatif est crédible, soutenu par une majorité au Parlement britannique Madame la secrétaire d'État, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être caractérisé de plan alternatif crédible ? Comment croire qu'un tel plan est encore possible, alors que cette dernière semaine nous a prouvé le contraire ? Ne serait-ce pas un risque de discrédit pour l'Union européenne que d'accepter un report long aux conséquences déstabilisatrices incertaines pour le fonctionnement de l'Union comme pour les élections européennes de mai ? Le Parlement britannique a dit « non » à un, « non » à une union douanière avec l'Union européenne, « non » à un maintien dans le marché unique, « non » à un second référendum sur l'accord de retrait. Tout se passe désormais comme si le bateau naviguait sans capitaine à son bord. Madame la secrétaire d'État, quelle position adoptera la France lors de ce sommet extraordinaire du 10 avril ? En dehors du Brexit, ce Conseil européen était aussi destiné à débattre d'une position commune face à la Chine, afin de préparer le sommet bilatéral Chine-Europe du 9 avril, sur fond de visite d'État du Président chinois à Rome, à Monaco et à Paris. Le défi est colossal, puisque jusqu'à présent l'Europe a surtout brillé par un manque de ténacité et un manque d'unité face à la Chine. Il ne s'agit pas de nier l'importance de la coopération sino-européenne ni de défaire ces relations. En effet, comme l'a rappelé le Président de la République lors de la conférence de presse conjointe avec le Président Xi Jinping et la Chancelière Angela Merkel, le 26 mars dernier, « le dialogue entre la Chine et l'Europe est devenu incontournable pour la définition des équilibres mondiaux, pour la préservation du multilatéralisme ». Aujourd'hui, il importe surtout que nous nous donnions les moyens d'une coopération équilibrée et exigeante, d'une coopération respectueuse des intérêts européens et adaptée aux réalités du monde. Nous devons nous donner les moyens d'une véritable cohésion entre États européens, car ce qui s'est passé dernièrement avec l'Italie ne peut que susciter des doutes néfastes et de l'inquiétude. À ce propos, notre groupe se félicite de la démarche inédite qu'a engagée le Président de la République en invitant Jean-Claude Juncker et Angela Merkel à une réunion commune avec le Président chinois. Un tel front uni est une manière de dire : « Nous sommes un État, certes, mais un État européen. » Aujourd'hui, une prise de conscience s'opère, et c'est plus que louable. Il y a, d'un côté, la Commission européenne, qui, avec son récent mémorandum, donne une impulsion à une posture plus ferme et plus réaliste, en exigeant un rééquilibrage dans les relations économiques avec l'Europe, plus de réciprocité dans l'accès aux marchés publics chinois, plus de transparence et moins de distorsions concernant les subventions d'État. Il y a, de l'autre côté, un Parlement européen inquiet des « menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l'Union » et qui exhorte les États européens à se coordonner. Cette inquiétude à l'égard de l'entreprise Huawei et de sa place dans le déploiement de la 5G en Europe n'est pas dénuée de fondement. Ce sujet appelle à beaucoup de prudence. Sur ce point, madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous dire comment la France accueille la communication de la Commission européenne portant sur une approche concertée en matière de sécurité des réseaux 5G ? la Commission appelle chaque État membre à réaliser une évaluation nationale des risques liés aux infrastructures des réseaux 5G d'ici à la fin du mois de juin. Comment le Gouvernement compte-t-il procéder pour opérer cette évaluation ? À nous, parlements nationaux, de nous saisir également de tous ces enjeux géostratégiques et de cybersécurité ; aux États, la responsabilité de contribuer à bâtir une cohésion européenne. N'ayons pas peur d'affirmer nos convictions, de bâtir une Union européenne solide et suffisamment protectrice. N'ayons pas peur d'affirmer nos valeurs européennes de démocratie, de liberté et de paix, tout comme nos intérêts européens

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, quelle que soit l'issue des négociations en cours à Londres ou à Bruxelles, quelles que soient les conditions de la sécession du Royaume-Uni, avec ou sans traité, avec ou sans accord commercial, au sein ou à l'extérieur de l'Union douanière, le moment que nous vivons est historique et nous devons nous interroger, en toute honnêteté, sur les conséquences de cette scission pour une Europe qui se questionnait, jusqu'à présent, sur les conditions de ses élargissements successifs. Il serait trop simple et trop commode d'expliquer ce repliement par l'isolationnisme atavique d'une nation insulaire ou, comme je l'ai entendu dans cette enceinte, par l'irrationalité d'un peuple et de sa classe politique offrant à une Europe sage et raisonnable le spectacle du « suicide d'une nation ». Je suis consterné aussi par les déclarations de celles et de ceux qui souhaitent que cette sortie de l'Union pénalise le peuple qui s'est détourné du droit chemin, et je déplore que le marasme attendu dissuade, à l'avenir, toutes nouvelles tentations de séparatisme. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de la situation que d'opposer aux Britanniques la fameuse formule d'une de ses dirigeantes : « Il n'y a pas d'alternative. M. Jean-Claude Juncker en propose une autre formulation quand il déclare : « Il ne peut y avoir de choix démocratiques contre les traités européens. » Dans l'esprit et la parole de ces contempteurs se déploie l'idée pernicieuse selon laquelle, finalement, le problème de la démocratie serait le peuple et que tout deviendrait plus simple et plus efficient si la politique était l'affaire des seuls spécialistes. Aux passions barbares et irrationnelles des multitudes incapables d'apprécier la justesse des moyens destinés à leur prospérité, il faudrait substituer le gouvernement des experts, détenteurs de la seule vérité et agissant pour le seul bien de l'humanité selon des règles économiques inspirées du seul bon sens. En comparaison, la rationalité d'un peuple est peut-être sommaire. Elle n'en repose pas moins sur la perception quotidienne de ses moyens d'existence, sur l'appréciation de ses conditions de vie et sur l'espoir d'offrir à ses enfants un monde meilleur. Tels étaient d'ailleurs les desseins constitutifs du traité de Rome de 1957. Je vous en rappelle deux motifs, Je vous en rappelle deux motifs, issus de son préambule : les États membres déclarent avoir pour but essentiel « l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples », et ils souhaitent « renforcer l'unité de leurs économies et en assurer le développement harmonieux, en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées Les États de 1957 formaient un ensemble relativement homogène par les niveaux de vie de leurs populations et les objectifs sociaux qu'ils s'étaient imposés au sortir de la guerre. L'élargissement de l'Europe à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal et à l'Irlande a été accompagné par des aides structurelles destinées à renforcer la cohésion économique et sociale de ce nouvel espace. Cette ambition a été abandonnée lors de l'adhésion des pays de l'est de l'Europe, alors même que leur situation économique et sociale aurait exigé un accroissement considérable de ces politiques de développement. Au contraire, dans ce nouvel ensemble très hétérogène, les disparités économiques et sociales ont entretenu des processus de mise en concurrence des individus, des entreprises et des territoires qui ont,, considérablement accru ces inégalités. Tout s'est passé comme si les mécanismes économiques déstabilisateurs inhérents au processus de la mondialisation avaient été introduits au sein de l'Union européenne. Soumises à ces pressions intérieures et extérieures, des régions entières de l'Europe ont subi un déclassement social et économique sans précédent ; ce sont leurs populations qui, au Royaume-Uni, ont voté massivement pour la sortie de l'Union. Ainsi, la rationalité du peuple britannique s'est exprimée pour condamner une dégradation de ses conditions d'existence, qu'elle attribue à l'Europe, parce qu'elle a bien perçu que sa logique économique obéissait aux mêmes dogmes que celle que leur avaient imposée les gouvernements de Margaret Thatcher. Le Président de la République a bien résumé cette profonde désaffection en déclarant, le 6 novembre 2018 : « Il faut entendre les peurs face à une Europe ultralibérale qui ne permet plus aux classes moyennes de bien vivre. Ce que nous disent aujourd'hui ces peuples qui se dressent contre l'Europe et dont nous devons absolument entendre les appels de détresse, c'est que les promesses du traité de Rome n'ont pas été tenues et que les engagements pris alors devant les nations ont été progressivement abandonnés. En réclamant le retour des frontières, ils souhaitent confusément que l'Europe, refondée sur son projet initial, organise notre espace commun sur d'autres règles que celles que tentent de nous imposer les États qui nous livrent une guerre commerciale totale. Nous ne pourrons poursuivre la construction de l'Europe contre les peuples. Les habitants de Stoke-on-Trent, près de Stafford, ont voté à plus de 60 % pour la sortie de l'Europe. Leurs raisons sont multiples, mais tous partagent le même désespoir devant la fermeture des dernières industries et le déclin inexorable de leur territoire. Il est grand temps d'entendre leur souffrance si nous voulons continuer à espérer dans l'Europe

le dernier Conseil européen s'est situé, beaucoup l'ont dit, dans le contexte du Brexit et des différents votes de la Chambre des communes. Ces votes, qui ont toujours

! Rappelons que les conséquences d'un Brexit dur ou d'un Brexit mou ne seront bonnes pour personne, pas plus pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni. Le Conseil des 21 et 22 mars a aussi été l'occasion d'aborder largement la croissance, l'emploi et la compétitivité. Approfondir l'Union économique et monétaire, mettre en oeuvre une politique industrielle volontariste, développer l'économie numérique ou encore se doter enfin d'une politique commerciale ambitieuse et protectrice : tels sont, avec les relations extérieures et le changement climatique, les principaux points qui Au-delà de ce qui peut apparaître comme un catalogue de bonnes intentions, on doit se féliciter du retour à une politique active et volontariste. L'Europe doit effectivement tracer des perspectives de développement, tout en assurant un haut niveau de protection. La Chine et les États-Unis sont, certes, des partenaires économiques de première importance, mais nous devons protéger nos entreprises de la concurrence déloyale de ces pays et leur permettre de se développer dans une économie désormais mondialisée.

On sortira alors des bonnes intentions pour entrer dans le concret, notamment avec des discussions concernant les perspectives budgétaires pour la période 2021-2027. Un nouveau Parlement européen aura été élu, et il sera temps

le Gouvernement assure qu'il fait tout pour maintenir son niveau au profit de notre pays. L'ancienne ministre, désormais candidate, a indiqué que la baisse pourrait être de 15 tandis que le ministre de l'agriculture parle, lui, d'au moins 5 %, mais il est dans son rôle. Peut-être pourriez-vous nous donner votre point de vue sur ce dossier majeur ? mes chers collègues. On en parle peu, mais il devrait nous inquiéter : il s'agit de l'avenir de la politique de cohésion. Cette politique est un marqueur fondamental pour l'Europe, car elle permet de réduire les écarts de richesse entre les pays de l'Union européenne, ainsi qu'entre les différents territoires au sein de ces pays. Or le flou le plus total règne sur le budget qui sera alloué dans le cadre financier pluriannuel ; et vous le savez, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup et qu'un mauvais coup se prépare ! Mme Loiseau, désormais candidate aux élections européennes, vient de déclarer qu'elle ne voulait plus que l'argent de l'Europe serve, à l'avenir, à construire des autoroutes en Slovaquie. C'est un peu désobligeant pour ce pays, mais c'est surtout inquiétant pour le nôtre. Nous voulons en effet, et je pense que nous serons tous d'accord dans cette assemblée, que l'argent de l'Europe continue de servir à construire des routes et à les aménager en France. Pour ma part, je trouve absurde d'opposer solidarité avec les territoires et compétitivité. L'une ne va pas sans l'autre, et il suffit de regarder le chemin parcouru par l'Espagne, le Portugal ou la Grèce pour se convaincre que l'aide apportée par l'Europe au développement, entre autres, d'infrastructures de transport

cas similaires : la première phase du désenclavement du bassin d'Alès, par la construction d'une 2x2 voies grâce à des fonds structurels, a permis à l'industrie de gagner en compétitivité et a attiré de nouvelles activités, notamment dans les services. Depuis maintenant plus de vingt ans, les conservateurs et libéraux n'ont eu de cesse que de vouloir modifier cette politique de cohésion, qui est une politique de solidarité, pour aller vers une politique de compétitivité.

pour les réformes structurelles qu'elle a proposé en mai 2018. Ce fonds contient d'ailleurs déjà une ligne réservée aux pays hors zone euro. Trois pistes de financement sont évoquées par la Commission, et c'est là que cela devient intéressant l'utilisation des 25 milliards d'euros déjà prévus pour ce fonds de soutien aux réformes structurelles ; le « refléchage » d'une partie des fonds européens prévus pour les 27 membres de l'Union européenne ; ou encore un prêt garanti par le budget européen. Ce projet a été discuté le 28 février et le 1 mars derniers par des représentants des ministères des finances des 19 pays, en même temps que la proposition franco-allemande sur le sujet. Dans ce document, les deux capitales conviennent de placer, comme le voulait Berlin, le budget de la zone euro au sein du cadre financier pluriannuel. Paris a obtenu, de son côté, que la gouvernance de cet instrument soit régie par un accord intergouvernemental. Le compromis contente les deux parties sur la nature des projets à cofinancer

Donc, si la proposition de la Commission européenne est approuvée, cela valide le principe d'une porosité des fonds vers les réformes structurelles qui seraient financées dans le cadre d'un budget de la zone euro. Je tiens à vous alerter tout particulièrement sur ce point, car, si on conjugue la conditionnalité des aides version allemande et Commission européenne à la création d'une enveloppe dédiée pour les pays de la zone euro, les fonds européens tels que nous les connaissons dans nos régions vont disparaître. Le groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen propose d'ailleurs le maintien et le développement de cette politique, si utile à nos territoires. De plus, le refus clair du Parlement européen, il y a quelques semaines, de l'application du principe de macro-conditionnalité doit être entendu et pris en compte. Nous l'avons déjà dit ici, voilà près d'un an, il n'est pas acceptable que la Commission européenne puisse intervenir au niveau des régions lorsqu'un État membre ne respecte pas les règles du pacte de stabilité et de croissance. Si nous validons dans le dur ce lien, cela ira irrémédiablement à l'encontre du développement de nos territoires, à l'échelle européenne. Madame la secrétaire d'État, la conditionnalité des aides, c'est faire payer aux citoyens européens les éventuelles turpitudes de leurs dirigeants, pour lesquels ils n'ont pas toujours voté. Pouvez-vous nous indiquer de manière claire et précise, si cela est aujourd'hui possible,

alors qu'il n'était pas initialement à l'ordre du jour du Conseil européen, le Brexit a naturellement accaparé la rencontre. Le terme du 29 mars est échu, et le Royaume-Uni n'est bien évidemment toujours pas sorti de l'Union européenne. Malgré la détermination de Theresa May, les différents accords n'ont pas été adoptés par le Parlement britannique, d'où cet allongement de délai. Dans ses conclusions, le Conseil européen a pris acte de la nouvelle échéance du 12 avril, un report que l'on ne peut qu'approuver sur le principe. Toutefois, le flou règne toujours, si ce n'est qu'en mettant sa démission dans la balance la Première ministre a quelque peu changé la donne. En attendant, la France et ses partenaires ne doivent pas relâcher leurs efforts pour parvenir à un accord de retrait, quitte à accepter un long report en respectant les deux conditions fixées par l'Union européenne, à savoir une participation des Britanniques aux prochaines élections européennes et un plan de renégociation clair.

c'est la seule alternative acceptable pour repousser la date du Brexit et ne pas risquer un désastreux. Nous connaissons en effet les enjeux de cette sortie dont nous examinons les contours depuis bientôt trois ans. Même si les États membres se préparent au pire des scénarios, comme notre pays l'a fait avec l'adoption d'une loi d'habilitation, est-on certain d'avoir cerné toutes les difficultés que pourrait engendrer la fin brutale d'une relation qui dure tout de même depuis Plusieurs millions de citoyens européens sont inquiets. Madame la secrétaire d'État, votre prédécesseur nous a apporté, le 14 mars dernier, quelques précisions sur la question de la circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Avez-vous aujourd'hui de nouveaux éléments de réponse sur le niveau des moyens de contrôle qui pourraient être rapidement mis en oeuvre aux frontières ferroviaires, maritimes et aériennes que nous partageons avec le Royaume-Uni ? le Royaume-Uni ? Au-delà de la sécurité technique et juridique du Brexit, la sortie du Royaume-Uni est bien entendu une affaire politique qui laissera des traces. Alors que des pays des Balkans se pressent aux portes de l'Europe, nous sommes en train de perdre l'une des plus anciennes démocraties parlementaires d'Europe, avec laquelle la France partage le même socle de valeurs, des valeurs qui nous poussent à bien des combats communs, par exemple en matière de sécurité et de défense. Je pense également aux accords de Lancaster House, pour lesquels plusieurs programmes sont en cours, notamment en matière de coopération dans le domaine des missiles. Si ces accords, de nature bilatérale, ne devraient théoriquement pas souffrir du Brexit, je m'interroge quant à la future place du Royaume-Uni dans la politique de sécurité et de défense. D'une façon plus globale, sans accord, que va-t-il advenir du cadre des relations futures entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, cadre que nous avions ébauché au travers de la « déclaration politique approuvée lors du sommet extraordinaire du 25 novembre 2018 ? Mes chers collègues, je veux être optimiste. J'appartiens à une formation pour laquelle la construction européenne demeure fondamentale malgré bien des aspects certes encore perfectibles. L'Europe s'est construite sur l'idée d'une paix partagée et, en cela, elle garde tout son sens. Comme l'a rappelé en forme d'adieu l'eurodéputé conservateur Richard Ash, « le Brexit représente un avertissement pour le peuple d'Europe. Nous ne devons jamais prendre pour acquis la paix prendre pour acquis la paix et la prospérité ». Aussi, dans cette perspective, l'Union européenne a encore de nombreux défis à relever. Il faut le faire Il faut le faire avec plus de célérité et plus d'audace ! Sur la crise financière, sur la crise migratoire, nous avons eu des réussites, mais les atermoiements et la lenteur des décisions ont ouvert la brèche à une contestation permanente de l'Europe par les partis populistes. Dans un monde plus ouvert, dans lequel de nouvelles puissances s'affirment et de grands ensembles se constituent, l'Union européenne doit conforter son projet. Il y va de nos souverainetés futures.

C'est une question d'équité et de justice fiscale. Je félicite en tous cas le Gouvernement français pour son volontarisme dans ce domaine. Sur le plan de la sécurité numérique, soyons vigilants sur la régulation de l'économie en ligne. C'est un sujet essentiel dont l'Europe doit se saisir dès maintenant, comme celui de la lutte contre la désinformation. Enfin, l'enjeu est de taille sur le dossier « Huawei Bruxelles souhaite « une démarche coordonnée de sécurisation des futurs réseaux 5G et " une évaluation " des fournisseurs de la future infrastructure ». Tout cela vous semble-t-il suffisant, madame la secrétaire d'État, alors que les États-Unis nous mettent en garde ? Mes chers collègues, à quelques semaines des élections européennes, bien que la question du Brexit hante les esprits, de nombreux dossiers méritent notre attention, tels que la PAC, la politique de défense et de sécurité, les enjeux d'innovation et de recherche, la politique industrielle. Notre engagement doit être total pour approfondir le projet européen et rappeler à nos concitoyens qu'il doit rester notre horizon. La

Mais il faut quand même le reconnaître : certains dirigeants européens, notamment M. Barnier, ont tout fait pour mettre de l'huile sur le feu.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat est l'occasion d'aborder le sommet Union européenne-Chine, sujet qui m'apparaît extrêmement important dans le contexte actuel. En effet, en quelques années, la Chine est devenue un acteur global, et plus seulement économique, une véritable puissance qui a su se construire patiemment, à bas bruit, au point d'être aujourd'hui omniprésente en Europe comme sur les autres continents. Le bras de fer économique entre les États-Unis et la Chine illustre combien, même pour l'hyperpuissance américaine, il est difficile de résister à l'avancée chinoise ou de trouver un terrain d'entente. Beaucoup découvrent, tantôt avec intérêt, tantôt avec stupeur, les tentaculaires nouvelles routes de la soie. Connues désormais sous le nom de, elles visent à bâtir des routes commerciales terrestres, ferroviaires, maritimes et numériques jusqu'à l'Europe, l'Afrique et plus loin encore. Ces différents projets, qui traversent de nombreux pays, mobilisent des milliards de dollars d'investissements dont la réalisation s'étale sur plusieurs décennies, bien qu'avançant à grands pas. Les conséquences économiques et géopolitiques de ce programme seront très importantes dans les prochaines années, d'autant que ces « routes » s'accompagnent d'un retour de la puissance militaire chinoise, destinée en partie à les sécuriser, c'est-à-dire à assurer la sécurité des ressortissants chinois et de leurs entreprises mobilisés en faveur de ces nombreux projets. Portée par les nouvelles routes de la soie et par une multitude d'accords bilatéraux, la Chine tisse un vaste réseau à travers le monde jusqu'en Europe, et même jusqu'à sa périphérie. Mais rien n'est le fait du hasard : qui se souciait du port du Pirée lorsque les Chinois en ont pris progressivement le contrôle ?

finalement, quel échec pour l'Europe de voir les PECO s'en remettre aux États-Unis et à l'OTAN pour leur sécurité, et à la Chine pour leur prospérité économique ! Par ailleurs, la Chine a constitué un véritable réseau d'organisations influentes à Bruxelles. Ces dernières agissent comme autant de leviers venant soutenir son effort diplomatique et sa stratégie de. tant qu'Européens, il nous faut donc être lucides dans l'analyse des événements et solidaires dans la réponse à y apporter. Je rappelle que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine et que 80 % des échanges commerciaux se font par voie maritime. des occasions sont à saisir : l'Union européenne devrait potentiellement profiter de cette augmentation des échanges dans les décennies qui viennent, à condition que cela fonctionne dans les deux sens, ce qui- vous le savez -n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Quant aux investissements chinois, ils sont en hausse en Europe, tandis que les investissements européens se sont réduits d'un quart en Chine. Il y a donc des rééquilibrages à faire. Puisque les routes maritimes, terrestres et ferroviaires vers la Chine existent désormais, quelle stratégie globale entendons-nous mettre en place pour favoriser l'export de produits européens dans ces conteneurs repartant vers l'Asie ? Quelles stratégies d'influence avons-nous en Chine ? Comment la France se donne-t-elle les moyens d'agir, quand d'autres pays semblent plus avancés ? De plus, si les investissements étrangers sont les bienvenus, les États ne doivent pas totalement se dessaisir de leurs infrastructures stratégiques. Une fois ces dernières cédées, tout retour en arrière serait difficile.

européenne ne devra pas se laisser instrumentaliser par Washington dans sa guerre commerciale avec Pékin. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à nous de voir si nous souhaitons être acteur du monde ou seulement spectateur de la compétition sino-américaine du XXI siècle ! Bravo ! Très bien

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2019. Le Royaume-Uni devait sortir de l'Union européenne le 29 mars dernier. Or il en est toujours membre ; mais jusqu'à quand, et sous quelle forme ? Lors du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019, les chefs d'État européens ont demandé aux dirigeants britanniques de se prononcer avant le 12 avril.

Notre territoire des Hauts-de-France, et plus spécifiquement le Pas-de-Calais, dont je suis l'élue, sera la victime toute désignée d'un Brexit dur. C'est sur cet enjeu que je centrerai mon propos, en complément de l'intervention de mon collègue Philippe Bonnecarrère. De nombreuses entreprises sont dépendantes de leurs échanges avec le Royaume-Uni. Pour illustrer l'importance de ces relations, nous pourrions évoquer les 31 milliards d'euros d'excédents que dégagent les exportations françaises vers le Royaume-Uni, et qui représentent 7 % du total de nos exportations. le secteur halieutique, 30 % de la pêche française se fait dans les eaux territoriales britanniques. Quant aux Britanniques, ils importent 42 % de leurs produits alimentaires depuis l'Union européenne. Mais, à l'heure actuelle, l'impréparation du côté britannique est telle que certains commencent à constituer des stocks pour anticiper les difficultés d'approvisionnement. Côté français, notre gouvernement a pris par ordonnances des mesures pour anticiper le et les entreprises ont été invitées à se préparer à leur échelle. Mais sont-elles réellement prêtes ? Le rétablissement des frontières douanières engendrerait des formalités administratives supplémentaires, un temps de passage portuaire accru, une désorganisation des chaînes logistiques et un coût supplémentaire, qu'il s'agisse du personnel ou de la formation.

Le maintien régulé des flux commerciaux, financiers et humains entre le Royaume-Uni et le continent européen, la pérennité des voies commerciales existantes sont cruciaux pour limiter les effets du Brexit sur l'activité économique et la mobilité de nos concitoyens.

cela soit bien clair pour tout le monde : les difficultés actuelles de blocages routiers côté français ne préfigurent en rien les possibles complications liées à la sortie du Royaume-Uni.

cet affaiblissement se ferait au bénéfice d'un transfert vers les ports du Benelux. Dans le cadre du Brexit, des mesures de contingence sont prêtes. Mais quand les déclencher ?

particulier à ses intérêts maritimes, parce que les secteurs du transport maritime, des ports européens, de l'industrie nautique et des énergies marines renouvelables sont des gisements d'emplois considérables, vecteurs de croissance et de compétitivité. l'indique le Président du Conseil européen, il est urgent de repenser les politiques commerciale et industrielle de l'Union pour faire face aux défis de long terme qui sont devant nous : dès lors, parions sur une stratégie maritime européenne intégrée En 2014, dans les sphères européennes, on parlait aussi d'une politique industrielle à l'ère de la mondialisation. La mondialisation des échanges passe aujourd'hui par les océans. s'agit donc d'une question éminemment européenne. Le 22 mars dernier, l'Union européenne a souligné : « Une base économique solide est d'une importance primordiale pour la prospérité et la compétitivité de l'Europe, ainsi que pour son rôle sur la scène mondiale. Cela appelle une approche intégrée tenant compte des défis actuels et émergents à l'échelle mondiale. » Au-delà des concepts, prenons le large : le volet maritime, s'il reste insuffisamment pris en compte, est au coeur des défis économiques de l'Union La Chine, devenue une puissance maritime de premier plan, l'a bien compris en prenant position dans divers ports mondiaux d'intérêt stratégique. Une politique industrielle volontariste repose aussi sur la maîtrise des espaces maritimes, avec le concours d'une marine océanique de premier plan. rappelé, l'Italie est le premier pays du G7 à entrer dans le projet des nouvelles routes de la soie. Un accord a été signé avec le Président chinois le 23 mars dernier. Les programmes d'investissements prévoient la modernisation des ports de Gênes de Trieste, qui deviendront les points d'entrée en Europe des routes commerciales maritimes. La France veut une nouvelle stratégie nationale portuaire : c'est utile, mais bien insuffisant si nous ne disposons pas d'une stratégie européenne portuaire commune à tous les États membres. Le document stratégique relatif aux orientations que la France souhaite donner aux politiques de l'Union européenne dans le domaine de la politique maritime au cours des cinq prochaines années doit être ambitieux. J'espère qu'il sera assorti d'un calendrier précis, avec des objectifs concrets.

le Royaume-Uni est le numéro 1 mondial de l'éolien offshore. Il entend ainsi renforcer sa position. Certes, cela nous fait réfléchir, mais le temps est à l'action pour développer sur nos côtes les énergies maritimes renouvelables, afin de combler notre retard. français CMA CGM et Ikea vont tester l'emploi de biocarburants sur un trajet au départ de Rotterdam de l'un des porte-conteneurs du groupe marseillais. C'est une initiative intéressante pour remplacer le fioul lourd. À l'heure où le fioul du navire souille l'océan Atlantique à proximité du littoral, avec une nappe d'hydrocarbures se déplaçant vers l'Espagne, il faut rappeler à l'Union européenne le rôle qu'elle doit jouer en matière de sécurité maritime, notamment depuis la création de l'espace européen de sécurité maritime, contenu dans le paquet « Erika III ». La création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en 2002, a été utile. Mais nous devons améliorer les dispositifs et le processus d'indemnisation. Le comité interministériel de la mer de 2018 indique l'importance des échanges de données entre secteurs du maritime et entre États membres de l'Union européenne. À la fin de 2019, la Commission doit présenter une une vision à long terme pour l'avenir industriel de l'Union européenne, assortie de mesures concrètes destinées à la mettre en oeuvre. Rappelons-lui que rien d'efficace ne se fera sans ambition maritime associée. dans son avis au roi : « La première chose qu'il faut faire est de se rendre puissant sur la mer, qui donne entrée à tous les États du monde. » Le XXI siècle sera maritime. L'Europe et la France doivent y prendre toute leur place : la tâche est donc immense ! Très bien

Ainsi, au vu des événements récents, dire que l'Europe avance en ordre dispersé face aux ambitions chinoises est un doux euphémisme. L'Italie a signé un accord séparé, d'ailleurs mal préparé et ne respectant pas forcément ses intérêts. Mais comment l'en blâmer si nous refusons de promouvoir et de mettre en place des champions industriels européens ? L'échec de la fusion d'Alstom et de Siemens ou encore notre incapacité à créer une alternative continentale dans le domaine de la 5G ne peuvent que nourrir les désillusions d'une Europe irresponsable et impuissante à servir ses propres desseins.

avenir. La réception du Président chinois à l'Élysée la semaine dernière, en présence de la Chancelière Angela Merkel et du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur invitation du Président de la République, va indéniablement dans le bon sens. Mais elle ne peut suffire à inverser le phénomène.

Ce sursaut européen est d'autant plus nécessaire que la Chine, quant à elle, se donne les moyens de ses ambitions. Les nouvelles routes de la soie soulèvent des enjeux majeurs et le financement pour les mettre en oeuvre atteint un niveau inégalé. La Chine a pour but de définir un nouvel ordre mondial dont nous devons être conscients. Avec mes collègues Pascal Allizard, Gisèle Jourda et Jean-Noël Guérini, nous avons détaillé ces enjeux dans un rapport publié l'année dernière. Les chiffres sont éloquents et donnent le vertige routes de la soie concernent directement plus de 70 % de la population, 75 % des ressources énergétiques et 55 % du PIB. Les montants consacrés par la Chine à cette politique atteindraient déjà 800 à 900 milliards de dollars. Ils seraient compris entre 5 000 et 8 000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. Les besoins de financement pour tous les projets rattachés aux nouvelles routes de la soie pourraient dépasser le trillion annuel un tel projet ne pourra être un succès, pour toutes les parties, que s'il fonctionne dans les deux sens. Pour ce faire, il est fondamental de créer les conditions d'un équilibre satisfaisant dans les relations entre la Chine, la France et l'Europe. Il convient de poser les bases d'un partenariat commercial fondé sur la réciprocité de l'ouverture des marchés, sur le respect de la concurrence, de la transparence et de la propriété intellectuelle, et d'un partenariat stratégique fondé sur une coopération multilatérale et cartellisée.

La cybersécurité, la défense, les frontières, le droit de la concurrence, le droit de l'innovation, le climat, ou encore le bouclier social : nous tous ici, moi la première, aimerions pouvoir faire avancer concrètement chacun de ces projets.

que l'Union européenne travaille bien sur les sujets concrets de la vie des Européens ; qu'elle apporte des réponses à un certain nombre de questions pour lesquelles les États membres, chacun avec ses prérogatives nationales, ne trouvent pas seuls les solutions.

de la politique de cohésion, il y a deux enjeux, et je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de politique ... Bien évidemment, nous aimerions conserver une politique de cohésion extrêmement ambitieuse-

si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, le nombre de sièges sera redistribué par pays de manière proportionnelle- cela signifie donc que la France aura plus de députés européens ; en revanche, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, ce sera le.

et la révision des règles européennes de concurrence. D'une part, le Conseil européen a invité la Commission à présenter, d'ici à la fin de l'année, une vision à long terme pour l'avenir industriel de l'Union européenne. Il l'a également priée d'élaborer, d'ici à mars 2020, un plan d'action à long terme visant à mieux mettre en oeuvre et faire respecter les règles du marché unique. Le Conseil européen demande, à cet égard, de mettre l'accent sur l'économie de services, notamment de données, d'approfondir l'union des marchés de capitaux et l'union de l'énergie- deux thèmes indissociables indissociables de la puissance de l'Union -et, enfin, d'assurer une fiscalité juste et efficace. Ces demandes du Conseil européen se situent dans une perspective plus globale, qui tend à conforter l'Europe comme une vraie puissance économique : cette stratégie d'ensemble intègre non seulement une politique industrielle volontariste et le marché unique, mais aussi l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, depuis une vingtaine d'années, profondément défaut, une politique numérique tournée vers l'avenir, et une politique commerciale ambitieuse garantissant concurrence loyale et réciprocité. Cette stratégie prometteuse me semble pouvoir constituer un socle valable pour la refondation de l'Union, à mener après les élections européennes. D'autre part, dans ses conclusions, le Conseil européen affirme la nécessité « d'assurer une concurrence loyale », non seulement « au sein du marché unique mais aussi « au niveau mondial », et « aussi bien pour protéger les consommateurs que pour favoriser la croissance économique et la compétitivité, conformément aux intérêts stratégiques à long terme de l'Union. Ces conclusions ont même été complétées pour préciser que l'Union européenne continuera d'adapter son cadre réglementaire « aux nouvelles évolutions technologiques et sur le marché mondial Le Conseil européen a également appelé la Commission à déterminer, avant la fin de l'année, les moyens de combler les lacunes du droit de l'Union européenne, afin de remédier, enfin, aux distorsions de concurrence induites par les entreprises étrangères lourdement subventionnées par leur État. Il a aussi évoqué la nécessité de revoir l'encadrement des aides d'État dans un sens propice à l'innovation. Les règles européennes de concurrence méritent effectivement un réexamen- le Sénat travaille depuis plusieurs années sur cette question en particulier. héritées de l'origine de la construction européenne, à l'heure où il s'agissait d'éviter les monopoles et ententes sur le charbon et l'acier, paraissent aujourd'hui totalement décalées.

Dans leur manifeste conjoint pour l'industrie, du 19 février dernier, les ministres français et allemand de l'économie envisagent l'introduction d'un pouvoir d'évocation du Conseil.

Le Sénat doit contribuer à cette réflexion essentielle ; c'est pourquoi la commission des affaires européennes vient de confier au groupe de suivi sur la stratégie industrielle de l'Union européenne, qu'elle a créé avec la commission des affaires économiques, le soin d'explorer la manière d'adapter les règles de concurrence, au service de l'ambition Cette ambition ne pourra pas se concrétiser si nous ne nous engageons pas davantage dans la numérisation de l'économie,

en matière de souveraineté numérique. Le Sénat travaillera également sur ce point. Ce sont donc des perspectives de moyen terme particulièrement importantes que le Conseil européen des 21 et 22 mars a tracées. À court terme, il devra reprendre rapidement la discussion sur trois sujets le changement climatique- question difficile -, la lutte contre la désinformation- c'est fondamental -, et le fameux dossier du Brexit. De fait, notre débat d'aujourd'hui se trouve faire aussi office de débat préalable au prochain Conseil européen. En effet,

et il faudra que, au travers d'accords bilatéraux, nous puissions trouver des moyens de convoler, ensemble mais différemment.

les mailles du filet entre la France et l'Allemagne. Cela repose sur un mot et un seul : la confiance, confiance de l'Allemagne vis-à-vis de la France dans ses politiques de réforme et dans sa rigueur budgétaire, confiance également de la France à l'égard de l'Allemagne, qui puisse un peu faire preuve de mouvement et d'innovation. Nous

La séance est reprise.

je suis naturellement très heureuse de vous présenter le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. En effet, ce texte revêt une importance particulière par rapport à l'action que ce gouvernement souhaite mener dans ses relations avec les territoires. Dans l'esprit du projet de révision constitutionnelle relative au droit à la différenciation, il s'agit de trouver des réponses institutionnelles adaptées aux besoins spécifiques des territoires. Il y a lieu non pas de provoquer un des compétences, mais d'ajuster ce qui peut l'être. En outre, sur la forme, ce projet de loi répond à une attente des départements alsaciens ; il est le résultat d'un processus de co-élaboration mené avec l'ensemble des parties prenantes et engagé l'été dernier. Nous venons en l'espèce accompagner une initiative locale. Voilà la méthode que je souhaite prôner : écouter, pour comprendre les aspirations des uns et des autres, et essayer de les concilier, en faisant du cousu main en fonction de l'expression d'une volonté territoriale. Depuis l'échec du référendum de 2013, qui visait à créer une collectivité territoriale unique regroupant le conseil régional d'Alsace ainsi que les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et depuis la création de la région Grand Est, l'Alsace n'a eu de cesse de revendiquer une évolution institutionnelle permettant de donner corps au « désir d'Alsace », tel qu'exprimé très majoritairement par la population. Une mission a été confiée au préfet de région Jean-Luc Marx en janvier 2018 pour mener une concertation sur la question institutionnelle alsacienne, sous deux réserves que la région Grand Est conserve son intégrité et que les grands équilibres actuels régissant les répartitions de compétences entre collectivités soient respectés. Le préfet a proposé d'opérer un rapprochement des deux départements au sein d'un nouveau département, lequel se verrait confier, dans le cadre du droit à la différenciation prévu dans la révision constitutionnelle, des compétences complémentaires essentielles au vu de son caractère transfrontalier très marqué.

Élisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, que je remercie vivement. Une déclaration commune engageant le Gouvernement, les deux conseils départementaux, ainsi que la région Grand Est a été conclue et signée le 29 octobre par le Premier ministre et les exécutifs des collectivités. Elle prévoit une réponse appropriée pour l'Alsace et trouve une part et trouve une part de sa traduction dans le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. La constitution de la Collectivité européenne d'Alsace se matérialisera par plusieurs étapes. Première étape, le regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en un seul département. Après que les deux conseils départementaux ont délibéré favorablement, à l'unanimité dans le Haut-Rhin et avec six voix contre dans le Bas-Rhin -, pour demander ce regroupement, le décret du 27 février 2019 a procédé à ce dernier pour constituer la Collectivité européenne d'Alsace. Deuxième étape, l'ajout- c'est l'objet du projet de loi que je vous présente aujourd'hui -de compétences particulières en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transports. le développement des politiques culturelles, économiques ou sportives dont les orientations étaient fixées dans la déclaration commune. Ces politiques font l'objet d'un travail approfondi avec les services déconcentrés de l'État et les autres échelons de collectivités concernées, et elles se traduiront, pour la plupart, dans des actes réglementaires. Le projet de loi s'attache à donner à l'Alsace des compétences suffisamment justifiées par ses spécificités pour que pour que le cadre constitutionnel actuel permette de les attribuer de façon pérenne et circonscrite à ce territoire. Il comporte des articles relatifs aux compétences- il s'agit des aux modalités relatives au personnel- articles 4 et 5 -, aux modalités de compensation des transferts- article 6 -, aux dispositions transitoires nécessaires au bon fonctionnement de la Collectivité de la Collectivité européenne d'Alsace- articles 7 et 8 -, aux ordonnances qui seront nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de cette collectivité, et aux ordonnances spécifiquement relatives au transfert des routes et permettant d'instaurer des « contributions spécifiques versées par les usagers concernés » aux termes de l'article 10. Au 1 janvier 2021,

Le projet de loi institue ainsi le principe d'un chef de filât de la collectivité, sur son territoire exclusivement, en matière de coopération transfrontalière. La collectivité pourra de ce fait organiser l'action collective, sans restreindre la capacité d'action des autres collectivités intéressées. également chargée d'établir un schéma alsacien de coopération transfrontalière, non prescriptif, en association avec l'ensemble des collectivités et des acteurs concernés. Elle aura, enfin, la capacité, en parfaite cohérence avec la stratégie régionale, de décliner un volet opérationnel sur les projets structurants en matière, par exemple, de santé, de mobilités, de formation professionnelle.

lieu, de compétences en matière de bilinguisme, pour renforcer ce vecteur culturel et ce facteur de mobilité professionnelle que constitue la langue allemande ; les Alsaciens ont beaucoup insisté sur la mobilité professionnelle. Les échanges que j'ai conduits, en lien avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, ont permis d'identifier deux volets particuliers pour développer l'enseignement de l'allemand d'abord, l'amélioration de l'attractivité pour les enseignants d'allemand titulaires recrutés par le ministère de l'éducation nationale, et,

afin de permettre l'enseignement de la langue au-delà des heures réglementaires, en complémentarité avec les programmes nationaux. La collectivité contribuera à la mobilisation d'un vivier pour que l'éducation nationale puisse accélérer les recrutements. L'éducation nationale lèvera les freins qui ont été identifiés ; l'État et la collectivité seront donc fermement engagés à obtenir, ensemble, des progrès à la hauteur des besoins.

en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Il s'agira, enfin, de compétences en matière d'infrastructures routières le projet de loi entérine le transfert, la gestion et l'exploitation des routes nationales et des autoroutes non concédées situées en Alsace, sur lesquelles, si elle le souhaite, la Collectivité européenne d'Alsace pourra lever des ressources spécifiques contribuant à maîtriser le trafic routier de marchandises- c'est l'objet de l'article 11. Il s'agit ainsi de régler définitivement un problème qui préoccupe les Alsaciens à juste titre et depuis longtemps. Par ailleurs, la Collectivité européenne d'Alsace pourra transférer à l'eurométropole de Strasbourg, sur sa demande, des portions de voies situées sur son territoire. Là encore, ce sont des sujets pour lesquels le Gouvernement a cherché à faire du sur-mesure pour l'Alsace, comme il souhaite pouvoir le pratiquer dans les territoires qui voudraient mener des projets dans une logique de différenciation. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi représente le point d'équilibre concret et pragmatique d'un processus d'élaboration avec les principaux intéressés. Je souhaite donc engager le débat qui va s'ouvrir en gardant une fidélité constante au processus politique qui a permis d'aboutir à la déclaration commune signée, le 29 octobre dernier, entre toutes les parties prenantes. Nous avons évité les écueils et nous sommes arrivés à un projet cohérent, qui permet de répondre au désir d'Alsace. Continuons sur cette voie ! La parole

l'histoire mouvementée de l'Alsace, ses particularités géographiques, son identité française et européenne, son bilinguisme ont largement fortifié l' qui justifie aujourd'hui la reconnaissance du « désir d'Alsace Cette spécificité alsacienne, régulièrement revendiquée, a été exacerbée par le redécoupage, en 2015, des grandes régions qui a totalement dissous l'Alsace dans la région Grand Est, et cela contre l'avis du Sénat. Mais c'est en 2018 que l'avenir institutionnel de l'Alsace s'accélère. Le 22 janvier, le Premier ministre, Édouard Philippe, lançait la réflexion sur le devenir institutionnel de l'Alsace au sein de la région Grand Est. Le 15 juin, le préfet Marx rendait sa copie en faveur de la fusion des deux départements, entité à laquelle pourraient être confiées des compétences nouvelles. Le 29 octobre, une déclaration commune était signée à Matignon, fruit d'une intense négociation entre le Gouvernement, les présidents des départements alsaciens- Frédéric Bierry pour le Bas-Rhin et Brigitte Klinkert pour le Haut-Rhin -et le président de la région Grand Est, Jean Rottner. Cet accord, ciselé à la virgule près, prévoit la création, au 1janvier 2021, de la Collectivité européenne d'Alsace, consacrant ainsi le regroupement des deux départements. Cette nouvelle collectivité doit bénéficier outre des compétences départementales, de prérogatives « particulières et supplémentaires », mais, à vrai dire, assez cosmétiques. Le 4 février dernier, les deux départements délibéraient pour demander leur fusion- à une très large majorité dans le Bas-Rhin et à l'unanimité dans le Haut-Rhin. Créée par le décret du 27 février 2019, cette nouvelle Collectivité européenne d'Alsace est donc bien un département. Tout juste ! Certes, un département « plus », mais pas plus que cela. Son nom baptismal, « Collectivité européenne d'Alsace », pouvait porter à confusion. C'est tout du moins ce qu'a considéré la commission des lois du Sénat, lui préférant l'appellation plus rigoureuse « département d'Alsace J'ai bien conscience que le nom « Collectivité européenne d'Alsace » est le fruit d'un subtil compromis, entériné par le décret qui prend acte de la fusion des deux départements et que le sujet de la dénomination est de l'ordre du symbole. Cependant, il ne doit pas cacher le coeur de nos débats, à savoir les nouvelles compétences de l'Alsace définies par le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui. Comme tout compromis, ce texte suscite de vives insatisfactions, tant de la part d'une partie des Alsaciens, qui souhaitent aller beaucoup plus loin, demandant même la sortie de la région Grand Est, voire la création d'une collectivité à statut particulier,

les difficultés provoquées par les deux réformes successives du redécoupage des régions et de la redéfinition des compétences régionales et départementales par la loi Cependant, même insatisfaisant, ce projet de loi est attendu par de nombreux élus alsaciens, car il donne du contenu à cette entité « Alsace » qu'ils appellent de leurs voeux les plus chers et dont ils ont très majoritairement décidé la création. Et si ce texte concerne principalement l'Alsace, il ne peut être déconnecté de la nécessaire évolution des lois de décentralisation, dont l'acte III est promis après la fin du grand débat national, ni de l'introduction dans la Constitution du futur droit à la différenciation, applicable à tous les départements français. La nouvelle Alsace doit être considérée comme une expérimentation dans la

collègues, je vous propose d'accepter le compromis négocié par les élus alsaciens et le Gouvernement et largement amélioré par le Sénat, afin non seulement de renforcer les compétences de la nouvelle Alsace et de lui donner les véritables moyens juridiques, humains et surtout financiers pour les exercer, d'expérimenter de nouvelles dispositions en Alsace qui auraient vocation à nourrir le débat général sur l'organisation territoriale de notre pays et à s'étendre aux départements qui le souhaitent et de sécuriser, dans la loi, les dispositions électorales initialement prévues par ordonnance. Concernant les compétences de l'Alsace, le texte initial prévoyait le transfert de prérogatives dans quatre domaines- coopération transfrontalière, bilinguisme, tourisme, routes nationales et autoroutes non concédées. Ces compétences ont une importance toute particulière en Alsace en raison des spécificités locales. La situation frontalière de l'Alsace et les liens privilégiés avec l'Allemagne justifient le développement d'une coopération transfrontalière affermie, notamment en matière de mobilité, d'échanges linguistiques, de coopération sanitaire la commission des lois a souhaité donner à la collectivité les véritables moyens pour les exercer. Chef de file, l'Alsace élaborera un schéma de coopération transfrontalière respectueux du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Elle pourra bénéficier de délégations des autres collectivités pour la réalisation des projets transfrontaliers, notamment en matière de déplacements. Afin de garantir son effectivité, le Sénat a autorisé les EPCI à déléguer tout ou partie de leur compétence à la nouvelle collectivité. Ces délégations seront essentielles pour mener à bien les projets de coopération transfrontalière en matière de transport et de mobilité des deux côtés de la frontière. Le développement des langues régionales et de l'apprentissage de l'allemand est primordial pour le développement économique et l'attractivité de l'Alsace frontalière. Ainsi, la collectivité alsacienne pourra organiser dans les établissements scolaires, sur le temps périscolaire, des activités complémentaires d'enseignement des langues et cultures régionales. De plus, elle pourra recruter un vivier d'enseignants germanophones et les mettre à disposition de l'éducation nationale pour favoriser l'ouverture de classes bilingues. Bien qu'inscrites dans la loi, ces dispositions restent programmatiques. Afin de les amplifier, la commission des lois a adopté les amendements de nos collègues alsaciens Reichardt, Kennel, Kern et Danesi confier à l'Alsace le chef de filât en matière de promotion des langues régionales et à étendre sa compétence à la formation des enseignants et à l'ouverture des classes bilingues ou d'immersion.

Conformément à la déclaration commune de Matignon, le Sénat a densifié la compétence du département d'Alsace en matière de promotion de l'attractivité de son territoire et prévu la création d'un conseil de développement tel que souhaité par le sénateur Kennel. Le transfert des 300 kilomètres de routes nationales et autoroutes non concédées à l'Alsace ne constitue pas véritablement une nouvelle compétence, puisque les départements gèrent déjà la majorité des voiries. L'innovation réside dans le transfert- pour la première fois -d'autoroutes à un département, ce qui se justifie par la nécessité de réguler le trafic provenant d'Allemagne, où la, la taxe sur les camions, favorise le déport de plus de 1 000 camions par jour sur les routes alsaciennes parallèles. Cependant, les conditions du transfert, telles que prévues par le texte initial, doivent être clarifiées, afin de donner à la nouvelle collectivité les véritables moyens pour endiguer la circulation des camions.

soumises aux règles applicables à la voirie départementale, et dont le déclassement pourra être décidé par le conseil départemental et sera nécessaire avant tout transfert à l'eurométropole de Strasbourg. La sécurisation du transfert des personnels affectés à la gestion et à l'entretien des voiries concernées est nécessaire pour éviter de se retrouver dans la situation de 2004, encore mal digérée par nombre de départements. Enfin, il convient de renforcer les garanties financières, afin de s'assurer que, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, le transfert de charges est réellement compensé par des ressources équivalentes. L'article 6 du projet de loi prévoit que les ressources attribuées

Enfin, elle a réintroduit dans le texte plusieurs dispositions électorales, afin de sécuriser ces procédures. Chers collègues, Alsaciens, élus du Grand Est ou du reste de la France, en adoptant ce projet de loi attendu par de nombreux Alsaciens, le Sénat remplira parfaitement son rôle de chambre des territoires. Entendant le « désir d'Alsace », la Haute Assemblée a souhaité amplifier les compétences reconnues au nouveau département fusionné, afin de lui donner les véritables moyens de les exercer. Mais le Sénat a aussi entendu la volonté légitime des autres départements de voir leurs spécificités territoriales reconnues au nom de la différenciation. C'est dans cet esprit que nous vous proposons d'adopter ce projet de loi, largement modifié.

madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues,

dont les identités territoriales ou régionales ont été malmenées, bafouées, niées, rayées de la carte, balayées du revers de la main par la création de grandes régions sur un coin de table, en une journée, à l'Élysée, sous la présidence de François Hollande. La question, c'est aussi celle du besoin de plus de décentralisation, de subsidiarité, de circuits courts dans les décisions publiques.

Le mouvement des « gilets jaunes » a révélé de façon éclatante cette crise de la démocratie représentative. Non que les représentants soient mauvais, mais ils ne sont pas écoutés. crise de la démocratie représentative, c'est d'abord une démocratie parlementaire entravée quand l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement et que le rôle du Sénat est contesté par l'exécutif. aussi une démocratie locale corsetée sur un plan réglementaire et étouffée sur un plan financier. C'est enfin une démocratie sociale bloquée qui n'a jamais bien fonctionné dans notre pays. pays. Montent des territoires un besoin de reconnaissance d'identité, de considération et une soif de libertés et de décentralisation.

depuis 1918, depuis notre retour à la France après une annexion qui avait, sur les plans administratif et universitaire, beaucoup plus pénalisé la Moselle que l'Alsace. Mais Paris a toujours davantage entendu les protestations bruyantes des Alsaciens que les pâles suppliques des Mosellans. ! Il n'y a de ma part aucune critique des Alsaciens, je leur dis même mon admiration. Ces revendications étaient légitimes et ils avaient le mérite de les porter plus fort. Aujourd'hui, ces justes revendications relayées par les Alsaciens sont partagées par tous les Français. Le Gouvernement ne peut satisfaire seulement ceux qui parlent plus fort en frustrant les autres. Cette inégalité de droit serait d'ailleurs anticonstitutionnelle. Satisfaire cette revendication dans un texte de portée générale exigerait, en l'état, au moins un renvoi à la commission.

parle des circonscriptions administratives de l'État, mais cela ne durera qu'un temps ... À une époque où l'État cherche à fermer le maximum de sous-préfectures et à regrouper les administrations techniques, Colmar ne restera pas préfecture éternellement

qui est constitutionnellement impossible. Certes, il existe en France métropolitaine, comme Paris et Lyon, des collectivités à statut particulier, mais reposant sur un critère démographique. De même pour la Corse, mais sur un critère physique- c'est une île

La Constitution ne permet pas une différenciation assise sur le critère culturel. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus de libertés pour les Alsaciens. Cela signifie qu'il en faut plus pour tout le monde.

par le bilinguisme et cette histoire singulière ; juridiquement, par le droit local ; géographiquement, par leur position frontalière et ces territoires étant l'un et l'autre traversés par un corridor européen nord-sud.

pourrait donc mettre en place une écotaxe poids lourds que le Gouvernement n'a pas souhaité permettre dans le projet de loi Mobilités que nous avons adopté cet après-midi même ! Or il nous faut l'écotaxe, que nos voisins allemands et suisses ont déjà instaurée, déviant ainsi tout le transit international nord-sud

En autorisant l'écotaxe en Alsace, et pas en Lorraine, le Gouvernement va provoquer le déport du trafic de l'A35 sur l'A31, réglant le problème sur l'A35, à la satisfaction des Alsaciens, mais l'aggravant d'autant sur l'A31, déjà à saturation, au détriment des Lorrains.

en raison des investissements sur les plateformes multimodales de Bettembourg au Luxembourg. La route de la soie arrive au port de Rotterdam. Elle se prolonge par le fer à Bettembourg. De là, les camions descendent par l'A31. C'est juste impossible

Cela suppose un texte de portée générale, respectueux des principes de la République. Ce n'est pas le cas de ce projet de loi, générateur d'inégalités et, à ce titre, anticonstitutionnel.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la présente motion vise à opposer l'exception irrecevabilité au projet de loi relatif aux compétences de la nouvelle collectivité territoriale réunissant les deux départements alsaciens. le raisonnement suivi par François Grosdidier, le texte prévoit d'accorder au nouveau département alsacien des compétences spécifiques de manière injustifiée et inopérante, d'une façon contraire à la Constitution.

Comme notre collègue le rappelle dans l'objet de sa motion, l'Alsace ne serait certainement pas le premier territoire à se voir doter de compétences dérogatoires du droit commun. Sans même avoir à porter nos regards vers l'outre-mer, la Corse, Paris et Lyon sont autant d'exemples métropolitains La Constitution laisse en effet au législateur une certaine latitude dans l'ajustement des missions et compétences des collectivités. Son article 34 le charge de déterminer les principes fondamentaux de « la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Et si l'article 72 prévoit que la loi peut créer des collectivités à statut particulier et toute autre collectivité territoriale, il n'exclut pas pour autant l'ajustement de certaines compétences des collectivités de droit commun, dont les départements. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans une décision de 1991, que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose pas au règlement différent de situations différentes, pour des raisons d'intérêt général. Absolument ! Certes, le choix du Gouvernement dans la présentation de son projet pour l'Alsace n'est pas le plus intuitif

Le processus législatif ne fait que commencer et ces points auront donc, si le législateur le juge utile, l'occasion d'être revus et corrigés. S'interdire de le faire dès le départ serait excessif. De même, si je comprends que l'on puisse regretter que la situation de l'Alsace ne soit pas discutée à l'aune d'une réforme plus globale des collectivités, l'absence d'une telle réforme n'interdit pas, sur le plan constitutionnel, une loi d'une portée plus limitée. Là encore, rejeter le simple examen du texte n'est pas la réponse la plus mesurée. Enfin, concernant les justifications concrètes des compétences différenciées du nouveau département, le transfert de compétences relatives au transport ne constitue pas une entorse à l'unité et à l'indivisibilité de la République. Compte tenu de la situation particulière du corridor rhénan, rhénan, principal axe de transport fluvial de notre continent, l'exercice de ces compétences sur le plan local mérite au moins d'être débattu. Je n'entends pas me prononcer ici pour ou contre cet aspect particulier des compétences de la collectivité alsacienne, mais je veux souligner qu'en discuter devant le Parlement est légitime et conforme à la Constitution. S'il faut en débattre, débattons-en ! Il s'ensuit qu'en adoptant aujourd'hui cette motion, nous courrons le risque d'écarter le Sénat de l'élaboration d'un texte important pour l'avenir de l'Alsace et des collectivités territoriales de l'Hexagone en général.

Il est préférable de prendre aujourd'hui le temps d'y travailler, de discuter de la forme de cette collectivité alsacienne et de faire entendre la voix du Sénat, au service de l'Alsace et de toutes nos collectivités. Pour ces raisons, je vous invite, mes chers

n'interdit pas au législateur de confier des compétences différentes à des collectivités territoriales appartenant à la même catégorie juridique, pourvu que ces différences soient justifiées par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général-

Monsieur le sénateur François Grosdidier, vous vous interrogez sur la constitutionnalité de l'octroi de compétences supplémentaires à la Collectivité européenne d'Alsace. Il s'agit d'un point de droit évidemment très important que le Gouvernement a pris pleinement en compte. Il a ainsi saisi le Conseil d'État de la question, à Constitution constante, de la différenciation de la répartition des compétences entre collectivités d'une même catégorie. Dans son avis du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a considéré que certaines différences dans la répartition des compétences étaient possibles, à condition de présenter un caractère restreint, dans les limites fixées par le principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a jugé, dans sa décision du 6 mai 1991 sur la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, que le principe constitutionnel d'égalité applicable aux collectivités territoriales « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». est précisément la situation de l'Alsace : les compétences supplémentaires que le projet de loi vise à confier à la Collectivité européenne d'Alsace sont justifiées par l'intérêt général et par la situation propre au territoire alsacien. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État l'a parfaitement reconnu en ce qui concerne la question des routes. Il a également estimé que les deux départements alsaciens étaient, en matière de langue et de culture régionales, dans une situation particulière. De manière générale, l'avis du Conseil d'État ne mentionne en aucune manière une inconstitutionnalité des compétences spécifiques qu'il s'agit d'attribuer à la Collectivité européenne d'Alsace.

vous considérez que rien ne s'oppose à ce que les autres départements frontaliers ou ceux qui sont fortement marqués culturellement bénéficient de compétences similaires à celles qui sont confiées à la Collectivité européenne d'Alsace. Vous vous demandez pourquoi la situation de ces autres départements n'est pas réglée dans le cadre de ce C'est pour une raison simple : le Gouvernement considère que l'exercice de compétences supplémentaires doit répondre à la demande et à la volonté des collectivités concernées.

j'ai beaucoup de sympathie pour les Alsaciens, singulièrement pour les sénateurs alsaciens. Pour autant, il arrive que, en certaines circonstances, je ne les rejoigne pas. Je leur rappellerai, s'agissant du « désir

Avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, le gouvernement Valls a accéléré la course au gigantisme par la fusion autoritaire des anciennes régions.

sur délibérations des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés, après consultation des populations concernées. En fait, l'augmentation de la taille des régions repose sur une erreur fondamentale, qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a d'économies d'échelle.

Compte tenu des frais de déplacement et de l'éloignement des centres de décision, les grandes régions n'ont donc permis aucune économie réelle de gestion. C'est ce que confirme un rapport de la Cour des comptes.

pour rien qui pourrait coûter cher. En fait, le cas de la région Grand Est et de l'ancienne région Alsace est particulièrement emblématique. En effet, la problématique d'une étendue territoriale démesurée s'y cumule avec celle de la disparition d'une ancienne région, l'Alsace, dont l'identité très forte est progressivement étouffée. La région Grand Est est deux fois plus grande que toute la Belgique, pourtant divisée en trois avec la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.

Il n'est donc pas étonnant que le quotidien du 18 juillet 2018 ait révélé une augmentation de 51 % des frais de déplacement et de mission de la région Grand Est en 2017 par rapport au total des trois anciennes régions en 2015. Et voilà ! Tout Et voilà ! Tout comme les Corses, la population alsacienne est très attachée à son territoire et à son identité. C'est le fruit de la géographie, de l'histoire et de spécificités aussi bien linguistiques que religieuses.

Dans la mesure où les Alsaciens sont presque unanimes à souhaiter le rétablissement de l'ancienne région, il est surprenant que le microcosme politique soit, lui, plus divisé sur le sujet.

ne veulent pas désavouer une réforme emblématique du gouvernement Valls. De leur côté, les élus LREM et MODEM s'alignent sur la position de l'actuel gouvernement et du locataire de l'Élysée.

Seulement, sans aucun scrupule, il a changé radicalement de position depuis qu'il a récemment été élu président de la région Grand Est. De nombreux vice-présidents du Grand Est réagissent de la même façon, motivés

Quoi qu'il en soit, le président Macron et son gouvernement sont parfaitement conscients de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Cependant, ils partagent la pensée dominante des cercles parisiens, selon lesquels plus une région est étendue, mieux elle fonctionne. Le Gouvernement craint aussi que la prise en compte de la demande alsacienne n'ouvre la boîte de Pandore des revendications territoriales d'autres régions. C'est la raison pour laquelle il s'oppose au rétablissement de l'ancienne région Alsace. revanche, afin de donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose une hypothétique alternative. Elle consiste à fusionner les deux départements alsaciens pour créer un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales. Selon son bon vouloir, la région Grand Est pourrait aussi lui déléguer quelques petites attributions. À l'évidence, cette Collectivité européenne d'Alsace n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun. Il s'agit par exemple du logo de l'Alsace sur les plaques minéralogiques. Avec cela, les Alsaciens iront loin De plus, et ce à juste titre, les autres départements de la région Grand Est ont d'ores et déjà indiqué que, s'il y avait délégation d'attributions régionales, ils demanderaient à bénéficier du même traitement, ce que M. Rottner et la région Grand Est refusent.

Quant aux territoires des deux autres anciennes régions, ils continueraient à être englués dans une région Grand Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. Manifestement, seuls le Gouvernement,

Face aux aspirations très fortes exprimées par les Alsaciens et aux problèmes inextricables que crée l'étendue démesurée de la région Grand Est, la seule vraie solution est de rétablir une région Alsace de plein exercice. Cela permettrait à la fois aux Alsaciens de retrouver leur identité et aux territoires des deux autres anciennes régions d'avoir de nouveau une gestion de proximité au plus près des réalités du terrain.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la présente motion, M. Masson invite la Haute Assemblée à opposer la question préalable au projet de loi relatif aux compétences de la nouvelle collectivité territoriale réunissant les deux départements alsaciens. Dans l'objet, il affirme que ce texte ne règle pas certains problèmes concernant l'étendue de la région Grand Est et ignore la volonté des Alsaciens de voir rétablir une région Alsace de plein exercice. Il est vrai, les changements de la carte des régions sous la mandature Hollande ont parfois pu causer des frustrations. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet dans d'autres contextes, car la taille de la région Grand Est et, de manière générale, le découpage des nouvelles régions ont été régulièrement critiqués. je ne pense pas qu'en examinant ce projet de loi le Sénat ignore la volonté des Alsaciens ni le désir d'Alsace manifesté par les citoyens et les élus alsaciens, bien au contraire ! si une hypothétique remise en cause de la structure de la région Grand Est n'est pas le sujet de ce texte, celui-ci entame néanmoins l'aménagement d'un ensemble alsacien, en cherchant à offrir un commencement de réponse à ce « désir d'Alsace Refuser de discuter ce commencement de réponse et le remettre à demain signifie ignorer une série de questions se posant dans l'immédiat. Celles-ci affectent le quotidien des Alsaciens, le fonctionnement de leur collectivité et des administrations territoriales, avec lesquelles ils interagissent. Refuser de discuter signifie ne pas prendre en compte l'attente légitime de réponses concrètes sur ces sujets. ailleurs, le décret mettant en place la nouvelle collectivité départementale alsacienne a déjà été pris, après consultation des conseils départementaux et du conseil régional concernés. Refuser d'examiner ce projet de loi aujourd'hui, c'est d'ores et déjà en dessaisir le Sénat et envoyer le signal qu'il a préféré ne rien faire et laisser la main à l'Assemblée nationale. Or l'un des rôles de notre assemblée est bien, selon les termes de l'article 24 de la Constitution, d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République. Très bien ! Procéder ainsi ne serait donc pas rendre justice à notre rôle constitutionnel. Même dans ce cadre aux options limitées, je pense que le Sénat se doit d'apporter sa contribution à la mise en place de l'Alsace de demain. Les débats sur le fond et sur la forme sont légitimes, et doivent avoir lieu. Car la question de l'Alsace ne cessera pas de se poser, même si le Sénat venait à refuser de discuter ce projet de loi. Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues,

Ce que dit l'auteur de la motion à propos de la création de la région Grand Est et de la volonté très forte des Alsaciens d'en sortir est vrai. Mais la politique est l'art du possible.

cela aurait eu le mérite de la clarté et de la simplicité. Les deux conseils départementaux ont donc accepté de négocier un contrat

car ce texte constitue malgré tout une avancée par rapport à la situation actuelle. Rien ne s'oppose à ce qu'on puisse aller plus loin dans les années à venir. Je vous invite par conséquent, mes

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues,

les élus alsaciens ont souhaité redonner une existence institutionnelle à leur territoire, doté d'une identité particulièrement forte, tant historique que linguistique et culturelle. Répondant à la demande formulée conjointement par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Gouvernement a décidé, par un décret du 27 février 2019, que ces deux départements seraient regroupés à la date du 1 janvier 2021 en un nouveau département prenant le nom de « Collectivité européenne d'Alsace avec des compétences particulières, justifiées par les spécificités locales, en plus des compétences départementales. Le présent projet de loi constitue l'aboutissement de cette démarche. Il vise à tirer les conséquences techniques du regroupement des deux départements alsaciens et tend à renforcer, dans une mesure plus ou moins large, les compétences du nouveau département alsacien dans les domaines de l'action transfrontalière, de la promotion des langues régionales, du tourisme et de la voirie routière. Néanmoins, l'ambition de ce texte demeure très modeste. La mesure la plus substantielle consiste en un transfert par l'État de l'intégralité de la voirie nationale non concédée à la nouvelle collectivité alsacienne, censé lui permettre de mieux maîtriser la circulation routière sur sur son territoire- cela a déjà été évoqué. Aussi, je me réjouis que la commission ait souhaité consolider les compétences de la nouvelle collectivité et lui donne les moyens humains, financiers et juridiques de les exercer.

Par ailleurs, en permettant aux EPCI à fiscalité propre de déléguer leurs compétences au département d'Alsace pour la mise en oeuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, la commission a entendu donner audit schéma une plus grande souplesse d'exécution, par par exemple en matière de mobilité. Concernant les langues régionales, je me félicite tout particulièrement que les attributions du département d'Alsace dans ce domaine aient été renforcées. La nouvelle entité serait ainsi désignée chef de file, sur son territoire, de la promotion de l'allemand standard et des dialectes alsaciens. Dans le même sens, la compétence des collectivités territoriales pour créer des chaînes de télévision en langue régionale a été consolidée. Je souhaite également souligner l'assouplissement de la répartition des compétences économiques. En effet, à titre expérimental, le conseil régional du Grand Est a été autorisé à déléguer tout ou partie de l'octroi d'aides aux entreprises au conseil départemental d'Alsace. Tout autre département pourrait demander à s'associer à cette expérimentation. Sans remettre en cause le rôle prééminent des régions en la matière, il s'agit d'introduire plus de souplesse dans la mise en oeuvre des politiques de développement économique, sur une base conventionnelle. En outre, la commission a souhaité garantir au nouveau département alsacien la compensation intégrale des charges nouvelles qui lui incomberont en raison du transfert de la voirie nationale non concédée, conformément à l'article 72-2 de la Constitution. Elle a donc intégré une partie des dépenses faites par l'État au titre du contrat de plan État-région à la base de calcul de la compensation financière, tout en offrant une garantie supplémentaire à la nouvelle collectivité en ce qui concerne les charges de fonctionnement et d'investissement de l'État qui seront prises en compte dans ce calcul. De même, la commission a renforcé la clause de sauvegarde relative aux emplois transférés par l'État. Enfin, elle a prévu l'institution d'un conseil de développement auprès du département alsacien, qui serait une instance de dialogue et de réflexion visant à accompagner la mise en oeuvre de ses compétences. Elle a aussi fixé dans la loi le nombre de cantons du département d'Alsace et adapté les règles relatives à l'élection des conseillers régionaux et des sénateurs de ce territoire. Madame la ministre, mes chers collègues, toujours très attentif au besoin de proximité qui s'exprime en Alsace, mais également sur l'ensemble du territoire, le groupe Les Indépendants votera ce texte ainsi modifié et surtout enrichi par la commission des lois.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, aujourd'hui, il est demandé au Sénat d'accompagner les Alsaciens et leurs élus dans leur volonté de donner une traduction institutionnelle au « désir d'Alsace » qu'ils portent dans leur coeur depuis toujours, et plus profondément encore depuis la refonte de la carte des régions en 2016. Cette volonté tenace traduit à la fois un attachement collectif et un projet commun attachement à une histoire, à une culture, à un patrimoine et à une mémoire communs ; projet de consolider un territoire transfrontalier ouvert sur l'Allemagne et la Suisse et de coconstruire un collectif capable d'agir avec proximité et efficacité en faveur de l'attractivité du territoire et de la vie quotidienne de ses habitants. Le projet de Collectivité européenne d'Alsace est réfléchi, construit, je dirais même qu'il est raisonnable. Pourtant, il attire des critiques. Pour les partisans de la sortie de l'Alsace de la région Grand Est, il ne serait qu'un leurre, un écran de fumée, une tromperie. Pour d'autres, en revanche, ce projet est une grave atteinte au principe d'indivisibilité de la République. Il faudrait donc interdire toute initiative locale émanant des territoires par peur d'une désintégration de la Nation au profit d'un repli sur soi frileux n'est pas ma conception de la République. Je trouve stérile d'opposer radicalement universalisme et particularisme. L'Alsace veut écrire une nouvelle page de son histoire en laissant plus de place à la diversité. Et, loin de se retrancher égoïstement sur son territoire, elle veut construire de nouvelles solidarités, notamment avec ses voisins européens. Pierre Pflimlin résumait ainsi le rapport de notre territoire avec nos voisins : « Je suis européen parce que je suis alsacien ». La Collectivité européenne d'Alsace s'inscrit également dans la continuité des engagements pris par le Président de la République en matière de relation avec les territoires : accompagner les initiatives dès lors qu'elles sont portées à l'échelon local et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt général, mais sans pour autant provoquer un big-bang des compétences. Je veux rappeler combien ce projet est le fruit d'un long travail de concertation entre le Gouvernement et l'ensemble des acteurs institutionnels, dont les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et le conseil régional du Grand Est.

Je salue également le rapport du préfet de la région Grand Est, Jean-Luc Marx, missionné en janvier 2018 pour évaluer les différentes hypothèses institutionnelles dans le respect des grands équilibres de la loi NOTRe. aussi remercier le Gouvernement, qui a entendu et soutenu ce « désir d'Alsace ». Madame la ministre, vous vous êtes rendue à de nombreuses reprises sur le terrain et avez travaillé en lien étroit avec vos collègues du Gouvernement, Élisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer. Les élus et le Gouvernement ont élaboré un projet institutionnel cousu main, avec la fusion des deux départements sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace », le socle de compétences départementales étant enrichi de compétences particulières

que nous allons examiner. Sous l'impulsion de Mme la rapporteure, la commission des lois a adopté plusieurs amendements visant à préciser, à approfondir ou à élargir les modalités d'exercice des compétences de la future collectivité. Ce sont là, pour l'essentiel, des avancées positives, que je tiens à saluer, avec quelques réserves de fond. Sans surprise, nous sommes plusieurs dans cette enceinte à souhaiter élargir encore le champ des possibles, en respectant les compétences des autres collectivités. Je souhaite, à titre personnel, que ces amendements « alsaciens » soient adoptés, afin que la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace soit la promesse heureuse d'un avenir serein. J'ai en revanche un point de désaccord profond avec la commission des lois au sujet du changement de nom de la future collectivité : pourquoi débaptiser à Paris la collectivité née en Alsace ? Je vous rappelle que l'appellation « Collectivité européenne d'Alsace » figure dans le décret du 27 février 2019, qui a procédé à la fusion des départements, ainsi que dans les délibérations des deux assemblées départementales adoptées le 4 février Au nom de quoi balayer d'un revers de main le fruit d'un accord patiemment construit ? Le Conseil d'État avait certes une préférence pour l'appellation « département d'Alsace », au motif que le nom « Collectivité européenne d'Alsace » serait susceptible de créer une méprise. Mais le Gouvernement et les deux départements ont tranché. Alors, de grâce, mes chers collègues, rétablissons la dénomination choisie ! Je vous le dis en toute franchise : imposer aux Alsaciens, en fin de parcours, un nom qu'ils n'ont pas choisi serait une marque de mépris qui affecterait longtemps l'image de notre assemblée. On tremble ! Sous cette sérieuse réserve, mon groupe votera pour l'adoption de ce projet de loi. Pour finir sur une note alsacienne, je formule le voeu que la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace trouve en notre assemblée la cigogne bienveillante qui livrera le nouveau-né à la maison. Car, comme le dit notre proverbe, quand les cigognes sont là, le monde est en bon état. « » Traduction : « Nous ne voulons pas une Alsace libre, mais une Alsace sereine.

Pardonnez-moi : je ne suis pas une cigogne ... Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au nom du droit à la différence territoriale, ce bricolage législatif, ni fait ni à faire, est une nouvelle étape de l'opération de démembrement de la République indivisible qui porte le nom de France. cette entreprise ancienne, la loi NOTRe a marqué un temps fort, sans aller cependant jusqu'à autoriser des fiscalités indirectes à la demande. En l'espèce, c'est le cas : on innove Cette différenciation est assortie, comme d'habitude, du désengagement de l'État : transfert au nouveau département alsacien des routes nationales qui n'ont pas encore été transférées, de l'enseignement des langues étrangères et des classes bilingues. Si ce projet de loi est un prélude à l'acte III de la décentralisation, on peut craindre la suite. Rapiécer un habit qui est usé avant même d'avoir été neuf n'est certainement pas la solution Quand on se penche sur les détails du texte, on va de surprise en surprise. Première surprise : il reprend le projet de fusion des deux départements alsaciens soumis sans succès à référendum il y a six ans. Revenir par la voie législative sur les décisions référendaires qui déplaisent devient une manie dans notre beau pays ! Deuxième surprise : sauf erreur de ma part, cette unique collectivité départementale d'Alsace devra cohabiter avec deux administrations territoriales de l'État. Curieuse innovation, curieuse simplification ! Troisième surprise : la législation actuelle permettant déjà de déployer la coopération internationale, on ne voit pas bien

La vraie solution permettant de concilier différenciation territoriale et unité nationale consiste à revenir à notre tradition administrative, qui a toujours su garantir la place des petites nations locales dans la grande nation nation : revenir, donc, sur un découpage régional dont personne ne veut, parce qu'il est incompatible avec les réalités des territoires, et revenir sur la répartition bureaucratique des compétences entre régions et départements, sur la suppression de la compétence générale des départements, sur les boursouflures qui ont complexifié la gestion complexifié la gestion locale en augmentant la dépense publique au lieu de la faire baisser- on attend toujours les 20 milliards d'euros d'économies qui avaient été annoncés ! Contrairement à ce qui se colporte, le jacobinisme français n'est pas qu'un centralisme c'est un étrange mélange de centralisme et de liberté locale qui fait de la France le pays où l'échelon territorial de proximité, la commune, dispose de l'autonomie la plus grande. À ceux qui en doutent, je conseille d'aller voir ce qui se passe en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pierre Grémion l'a montré il y a bien longtemps : dans le système administratif classique, le préfet et son administration ne sont pas que la courroie de transmission de l'État central ; ils sont aussi les porte-parole des territoires et de leurs élus auprès de l'État,

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983, puis celles qui sont relatives à la coopération intercommunale volontaire de projet, à partir de 1992, viendront renforcer ce « pouvoir périphérique », pour reprendre l'expression de Pierre Grémion. C'est cet édifice administratif solide et efficace que les réformes des quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron ont voulu démonter, alors que c'est le contraire qu'il aurait fallu faire. En l'espèce, respecter la spécificité alsacienne passe non pas par la création d'une collectivité à usage particulier, mais par un redécoupage régional permettant de garantir un tel respect, ce qui est déjà possible dans l'état actuel de la législation. J'ai cru d'ailleurs comprendre que telle était aussi la position de bon nombre de collègues alsaciens. Selon Jérôme Fourquet, la France serait devenue un archipel d'îles et d'îlots sans liens entre eux, une nation multiple et divisée, autant dire autre chose qu'une nation. N'entendant pas participer à cette entreprise de destruction de l'unité nationale, le groupe CRCE votera contre ce projet de loi ni fait ni à faire, mais bien révélateur des intentions de ses auteurs.

Harribey. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, ce projet de loi constitue un prolongement logique du décret du 27 février 2019, qui crée le département d'Alsace en fusionnant les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Mais, en réalité, les auteurs de ce texte poursuivent deux objectifs procéder aux adaptations législatives rendues nécessaires par la fusion et tenter, par des articles à la formulation quelque peu alambiquée, de résoudre la question du statut institutionnel alsacien. nous, ce dernier volet relève davantage de la communication que du droit, et ne satisfait visiblement personne. Les débats en commission ont bien montré que c'était là la question prédominante.

l'échec du référendum d'avril 2013 sur la création d'une collectivité territoriale d'Alsace, en raison d'une trop faible participation et d'un vote négatif du Haut-Rhin ; le traumatisme causé par la création de la région Grand Est

en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Cette nouvelle entité vise, dit-on, à donner corps au « désir d'Alsace ». D'où le caractère dual de ce texte : d'un côté, un volet classique, qui vise à traduire en droit des évolutions institutionnelles ; de l'autre, l'objet est, donc, de donner corps à une nouvelle collectivité qui, fondée sur le socle des compétences départementales, devrait être enrichie de compétences supplémentaires et particulières, mais sans fondement juridique clair. clair. Le risque est de tromper les citoyens- les débats le montrent bien -, ... Eh oui ! ... puisqu'il ne s'agit en rien d'une communauté nouvelle à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, mais bien d'un département unique issu de la fusion de deux départements. En ce sens, le texte tel qu'il est présenté en séance clarifie les choses, la commission ayant adopté sur notre initiative la dénomination « département d'Alsace ». Par cette modification, la commission a simplement mis le texte en conformité avec la réalité. revanche, dans le cadre de cette discussion générale, nous voudrions mettre l'accent sur une autre question soulevée par ce texte : celle de la coopération transfrontalière qui touche non seulement l'Alsace, mais toutes les régions transfrontalières.

sans caractère prescriptif ni décisionnel qui s'ajouterait aux schémas existants élaborés à l'échelle de la région et de l'eurométropole. Mme la ministre a même précisé qu'il fallait que ce schéma soit « conforme En l'état, nous pensons que ce point reste insuffisamment défini et que le texte ne va pas assez loin. À l'article 13 du traité d'Aix-la-Chapelle, qui n'est certes pas encore ratifié, est pourtant

on peut certes regretter que ce projet de loi ait été vu comme une opportunité de faire croire que la collectivité d'Alsace allait bénéficier d'un nouveau statut, mais l'essentiel, selon nous, a été corrigé avec le changement de dénomination.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, à peine quatre ans après l'adoption de la loi NOTRe et le redécoupage à la hache des régions, nous sommes amenés à débattre aujourd'hui d'une des premières conséquences de cette nouvelle organisation territoriale, que beaucoup ont à juste titre qualifiée de « mariage forcé Bien sûr, nous sommes avant tout des républicains, respectueux de la légalité et de la souveraineté exprimées par le Parlement. La loi doit être appliquée en toutes circonstances, même si nous sommes réduits à compenser des erreurs originelles. En deux ans, les nouvelles régions n'ont pas ménagé leurs efforts pour relever de nouveaux défis et tâcher de satisfaire l'intérêt général. Mais, en tant que législateurs, notre devoir est d'examiner le présent projet de loi à l'aune de deux principes qui nous sont chers le caractère un et indivisible de notre République décentralisée, d'une part, et l'égalité entre tous les citoyens, d'autre part. Certes, un « désir d'Alsace » s'est fortement exprimé depuis 2015. Le Président de la République, tout en réaffirmant que le Grand Est ne serait pas détricoté, a voulu que se noue un dialogue qui a conduit à un accord entre l'État, la région et les deux départements alsaciens. Cet accord prévoit donc la fusion des deux départements au sein d'une nouvelle collectivité, et le transfert de certaines compétences : coopération transfrontalière, bilinguisme, routes et tourisme. Nous ne sommes pas opposés par principe à la fusion des deux départements alsaciens, dès lors qu'elle correspond à une volonté clairement exprimée et qu'elle est accompagnée de garde-fous correspondant aux principes que j'ai rappelés. Mais nous nous interrogeons- je ne vous le cache pas -sur l'opportunité de légiférer dès maintenant sur le cas alsacien, alors même que la réforme constitutionnelle, toujours en navette, doit précisément prévoir les conditions d'un droit à la différenciation des collectivités. Pourquoi l'Alsace aujourd'hui, alors que le régionalisme parvient à s'exprimer par de multiples voies dans notre pays ? Pourquoi, en outre, ne pas donner la priorité aux territoires les plus en difficulté ? Je vous rappelle également que le Conseil d'État a émis des réserves, craignant que cette fusion ne crée des doublons, alors que nous avons en tête l'exemple des conséquences des fusions de régions. Certains arguments invoqués pour justifier la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin me semblent par ailleurs caducs, comme la nécessité de pouvoir dialoguer d'égal à égal avec les Länder allemands il s'agit précisément du rôle de la région Grand Est, car son poids le permet, sans compter que la Moselle est tout aussi concernée par ces questions du fait de sa frontière avec l'Allemagne.

la mobilité et au travail transfrontaliers. Le bilinguisme est également un sujet essentiel qui mériterait d'être développé dans toutes les régions frontalières. Et en quoi le périmètre le plus opportun serait-il celui de la nouvelle collectivité lorsque l'on parle numérique, culture ou transports ?

cet enjeu dans le périmètre d'une seule collectivité est à l'opposé de la vision à 360 degrés, ouverte à l'ensemble de la société, qui devrait être celle d'une République une, indivisible et décentralisée, particulièrement au moment où nos concitoyens expriment un besoin très vif de proximité. S'agissant du transport, parmi les questions régulièrement soulevées par nos concitoyens figure le passage des poids lourds étrangers sur les axes français et leur non-participation au financement des infrastructures sur notre territoire. Ce sujet a été évoqué au cours de la discussion du projet Aucune solution n'a pour l'heure été trouvée, et le Gouvernement nous a renvoyés aux conclusions du grand débat. C'est en partie cette raison qui justifie le transfert à la nouvelle collectivité des routes nationales et des autoroutes non concédées du domaine public routier national. Nous doutons que ce transfert puisse régler tous les problèmes, mais nous soutiendrons bien sûr l'ambition des élus locaux de lever de nouvelles ressources pour financer les infrastructures de transport et toutes les formes de mobilité.

étape vers un nouvel acte de la décentralisation, très attendu par les élus locaux. Le groupe du RDSE y est bien sûr très favorable et apportera sa contribution à ces travaux. Nous espérons toutefois que ce texte n'ouvrira pas la porte à une sortie de l'Alsace de la grande région. Et nous déplorons que la question de l'Alsace soit tranchée dès aujourd'hui, alors que la décentralisation sera au coeur des débats sur le projet de révision constitutionnelle. Ces réserves ayant été soulignées, le groupe du RDSE attendra les débats, qui ne manqueront pas d'être riches, pour se déterminer.